La séance est reprise et la parole est à madame Jocelyne Guidez pour une mise au point sur un vote. Merci madame la présidente. En effet je souhaiterais modifié mon vote, ainsi que celui de Madame, Denise Saint-Pé sur le scrutin numéro 97 sur la proposition de loi, droits de l'enfant du jeudi 8 décembre en abstention au lieu du vote contre.--

en situation de handicap ainsi que des assistants d'éducation dans l'action générale. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes âgées.-- Personnes âgées c'est un. J'en parlerai à mon psy. Ces personnes handicapées. Madame la présidente.-- Monsieur le président de la commission de la culture de l'éducation et de la communication. Madame la rapporteure.-- Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs.-- l'heure je m'exprime devant vous. Ce sont 430.000 élèves en situation de handicap. Qui sont scolarisés.-- À l'école de la République. Dans des classes dites ordinaires.-- Leur effectif. Connaissent une croissance de 6 à 10% par an.-- C'est avant toute chose. Une grande source de satisfaction. Pour ses enfants d'abord.-- Qui sont bien à la place qui est la leur, c'est-à-dire sur les bancs d'une école.-- Mais aussi pour celles et ceux qui accompagnent ses enfants. Et travaille avec eux à construire leur autonomie.-- Et cette, enfin je crois une. Réussite due à la mobilisation de tous. Et de l'État particulièrement depuis plus de 17 ans. C'est-à-dire depuis le vote de la loi du 11 février 2005.-- Et c'est bel et bien la mise en place d'une école inclusive telle qu'elle a été voulue par le président de la République. Et mis en place lors de son premier quinquennat.-- Le gouvernement engage aujourd'hui des moyens importants et croissants pour accueillir les élèves en situation de handicap dans de bonnes conditions.-- Il mobilise plus de 132.000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Les AESH.-- 4000 nouveaux AESH ont été recrutés à la rentrée 2022 et 4000 de plus sont prévus dans le projet de loi de finances pour 2023.-- Le nombre des AESH est ainsi en augmentation constante. Il a augmenté de 50% entre 2017 et 2022. Il y a aujourd'hui un AESH pour enseignants.-- Ce qui fait de ce métier. Le 2ème métier de l'éducation nationale en terme d'effectifs.-- Il faut prendre la mesure de ce que signifie une telle évolution. C'est précisément la philosophie de la proposition de loi discutée aujourd'hui qui entend contribuer à l'amélioration du système d'inclusion scolaire en renforçant la stabilité professionnel des accompagnants et accompagnante des élèves en situation de handicap.-- L'enjeu de ce texte est simple, madame la rapporteure, vous le savez. Il s'agit de rendre ce métier plus attractif en faisant en sorte qu'il ne soit. Plus un métier précaire.-- Je vous le dis sans détour, je partage avec vous tous, cette ambition.-- Et avant d'en venir à votre proposition, je tiens à rappeler que cette préoccupation s'est traduite dans les actes depuis 2017.-- Où de nombreuses mesures ont été mises en place pour améliorer l'attractivité du métier d'AESH et de ses conditions d'exercice.-- Le recrutement en CDD d'une durée minimale de 3 ans. L'accès au CDI au bout de six ans d'exercice. La mise en place d'une formation de prise de poste de 60 heures. L'accès aux droits à formation professionnelle et aux prestations d'action sociale.-- La création d'une grille indiciaire afin d'automatiser leur avancement. Et enfin la création de la fonction de référent à ESH. Afin d'appuyer leur exercice professionnel par des pairs expérimentés.-- Le gouvernement entend aujourd'hui poursuivre dans cette politique continue de consolidation de ces emplois, en prenant des mesures, des mesures fortes sur leur rémunération. Dans le cadre des crédits de la mission enseignement scolaire que vous avez adopté la semaine dernière, le gouvernement a soutenu des amendements qui permettront une augmentation salariale nette de 10% de tous les AESH dès le 1er septembre 2023. Une enveloppe supplémentaire de 80 millions d'euros sera ainsi consacré à cette revalorisation en 2023. Cette revalorisation s'ajoutera. À l'extension aux AESH. Et aux à ED. De la prime Rep et Rep Prévue par le projet de loi de finances et qui correspond à une enveloppe de 74 millions d'euros. Si ces mesures sont adoptées définitivement. Nous serons également en capacité de renforcer notablement l'investissement de l'État dans la formation de ces personnels. Sujet sur lequel je sais. Que le Sénat est particulièrement attentif.-- Les dispositions prévues par votre proposition de loi. Permette de poursuivre cette avancée.-- D'une part la situation sociale des AESH. S'améliorera le contrat à durée indéterminée présente l'Avantage de sécuriser les personnes dans leur emploi. Grâce à cette proposition. Les AESH seront désormais auront après un contrat de 3 ans. Contre 6 ans actuellement.-- Ce qui était effectivement trop long pour la perspective de stabilité que nous leur devons.-- D'autre part, cette amélioration des conditions d'emploi rendra ce métier plus attractif. C'est déterminant à un moment où nous rencontrons des difficultés à recruter et à fidéliser dans ce métier essentiel à l'autonomie des élèves en situation de handicap.-- C'est un progrès qui est réel qui est concret. Qui est applicable applicables rapidement sur le terrain et qui surtout est attendu par les personnes concernées.-- Par ailleurs, je tiens à apporter une précision supplémentaire. Concernant les dispositions prévues initialement pour lutter contre la précarité des assistants d'éducation. Est maintenu dans le texte que nous examinons aujourd'hui. Je veux vous dire et qu'elles le sont d'ores et déjà satisfaite. En effet, la loi de lutte contre le harcèlement scolaire. Adopté le 2 mars 2022 prévoit déjà un CDI obligatoire pour les à ED au bout de six ans et le décret qui en prévoit les modalités a été publié le 9 août 2022. Compte tenu de sa date de publication. Il n'a pas pu encore produire tous ses effets au moment de la rentrée 2022, mais ce sera bien le cas à la prochaine rentrée. En outre, la prime Rep et Rep plus leur est également adoptée dans le projet de loi de finances.-- Je veux donc pour conclure. Revenir sur la question des modes d'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école. Pour rappeler que l'aide humaine que constituent les AESH doit être inscrite dans un cadre plus large. Des élèves en situation de handicap doivent être scolarisés. C'est un droit, ce n'est pas une option.-- Et nous devons leur fournir les moyens d'accompagnement adéquates pour que notre école soit pleinement inclusive. Les AESH sont à cet égard des personnels essentiels irremplaçable pour notre école pour tous. nous entendons bien l'affirmer haut et fort on travaillant à améliorer leurs conditions d'exercice de ce métier. Mais il faut rappeler aussi l'esprit de la loi de 2005. Avec cette idée cardinale de l'adaptation à chaque situation de handicap. Or, tous les élèves n'ont pas besoin du même type d'aide pour apprendre et pour progresser vers l'autonomie. En outre, parmi celles et ceux qui en ont besoin. Tous n'ont pas besoin d'un accompagnement individuel. Par conséquent. La croissance continue du nombre d'AESH. Ne peut pas et ne doit pas être la seule réponse aux besoins d'accompagnement des élèves à l'école. Il est nécessaire de progresser sur les autres moyens d'accompagner efficacement les élèves en fonction de leurs besoins, notamment par exemple par l'usage d'outils numériques et notamment aussi à travers l'évolution des méthodes pédagogiques et de la formation des enseignants. Il faut aussi que nous avancions sur l'organisation administrative pertinentes pour conduire cette politique.-- C'est dans cette optique que s'est ouverte dans la foulée de la conférence interministériel du handicap du 6 octobre dernier, une phase de concertation et de réflexion avec les acteurs de l'école inclusive. Cette réflexion associe bien sûr les départements et les maisons départementales pour les personnes handicapées car il est nécessaire de repenser l'ensemble du processus d'évaluation des besoins des élèves et de notification des aides nécessaires. Cette concertation à laquelle des parlementaires sont associés aboutira dans le cadre de la conférence nationale du handicap que le président de la République convoquera au printemps 2023.-- Je veux redire pour terminer. Que la stabilité professionnel des accompagnants des élèves en situation de handicap ainsi que leur conditions de revenus sont déterminantes pour la qualité et l'effectivité de la scolarisation des enfants en situation de handicap. De cela dépend aussi l'attractivité de leur métier et donc sa pérennité agir et donc essentiel pour le bien-être de ses personnels mais aussi bien sûr pour celui des élèves. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement est donc favorable à cette proposition de loi, je vous remercie.-- Madame la présidente Madame la Ministre, Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. C'est la 2ème fois en l'espace de quelques mois que notre commission se penche sur la situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap personnel, cheville ouvrière de l'école inclusive en février avec mes collègues Annick Billon et Max Brisson. Dans le cas de la mission d'information que nous avons menées sur le bilan des mesures éducatives du précédent quinquennat nous lancions une première alerte sur leur conditions d'emploi et de travail aujourd'hui l'examen de cette proposition de loi dont je salue l'auteur ancienne députée Michèle Victory nous offre l'opportunité de tirer une seconde fois la sonnette d'alarme, mais aussi et surtout de faire avancer la législation reconnaissons d'emblée que la situation des 132.000 AESH, donc 93% 93% sont des femmes n'est pas acceptable ni digne de l'école de la République. Un mot suffit à les caractériser précarité, précarité que notre collègue Max Brisson ah lors de l'examen de la proposition de loi en commission très justement qualifiée d'institutionnaliser les causes et les manifestations de cette précarité sont nombreuses, d'abord les conditions de recrutement, plus de 80% des ASH exerce dans le cas d'un CDD, contre moins de 20% en CDI ensuite les conditions d'emploi, seulement 2% des AESH dispose d'un emploi à temps complet. La quantité de travail moyenne n'étant que de 62%. Ce temps hein combler subi contraint les AESH accumuler d'autres petits contrats pour prétendre à un niveau de revenu plus décent des conditions de rémunération précisément sous l'effet cumulatif du temps incomplet imposé d'une grille indiciaire concentré à des niveaux proches du SMIC. La rémunération mensuelle moyenne de et ça, je n'ai que de 850 euros Net l'état rémunère donc en dessous du seuil de pauvreté. Ces professionnels de l'école inclusive. Les conditions de formation, enfin dans les lacunes, tant à la prise de poste qu'en cours d'exercice laisse souvent les AESH démunis lorsqu'ils ne sont pas contraints de s'auto former à ce cumul de précarité viennent s'ajouter des conditions de travail qui de l'avis unanime des AESH mais aussi d'autres acteurs de l'école inclusive n'ont cessé de se dégrader depuis quelques années. La généralisation des pôles inclusifs d'accompagnement localiser des pial a assurément marqué un tournant dans leur aggravation au regard du premier bilan que Jean dresse dans mon rapport 3 correctifs me paraissent devoir rapidement être apportées, mettre un terme aux dérives d'une gestion de la ressource humaine basée sur la flexibilité. Replacer la qualité de l'accompagnement au coeur du dispositif renforcé le cadrage national pour assurer plus d'harmonisation entre les territoires aujourd'hui être à ESH sous fonctionnement de pial c'est être soumis à une très grande flexibilité affectation dans plusieurs établissements, ce qui entraîne de nombreux déplacements dans les frais ne sont pas toujours prises en charge changements fréquents et non concertée d'emploi du temps et d'affectation. Prise en charge simultanée de plusieurs enfants accomplissement de tâches, ne faisant pas partie d'émission, droit à la pause méridienne Méridienne et au fractionnement des jours de congé non respectés. Je me dois d'illustrer ce tableau pour le moins édifiant par les mots des intéressés eux-mêmes des conditions de travail déshumanisé, a-t-on entendu sentiment d'être du sous-personnel à ESH sous-payés et corvéables à ESH toujours relégué en dernier malgré l'absence de reconnaissance et la perte de sens, que ces professionnels dénoncent nombres d'entre eux ont le courage de continuer. Qu'est-ce qui les fait tenir la réponse tient en 2 citations à ESH c'est un beau métier sont-ils dit sans à ESH, il n'y a pas d'école inclusive. Alors que le métier d'AESH n'a jamais été aussi peu attractif. Le paradoxe veut que dans le même temps, les besoins d'accompagnement des élèves en situation de handicap croissent à une vitesse très soutenu. Depuis 2017 les notifications d'aide humaine Des MDPH augmente de 11% par an, soit à un rythme près de 2 fois supérieur à celui des notifications de reconnaissance du handicap. Cette tendance à la systématisation de l'aide humaine est un sujet qui appelle une réflexion conjointe de l'éducation nationale et des départements. Plus largement nos échanges en commission, ont montré que la prise en charge de l'enfant dans sa globalité. À la fois sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire, pose la question du partage des responsabilités. Notre commission entend bien l'approfondir. Dans le cadre de ses prochains travaux de contrôle. Bien que les effectifs d'AESH et progressé de 35% sur les 5 dernières années et qu'il continue d'augmenter. L'école inclusive n'a pas n'est pas encore une réalité pour tous les élèves en situation de handicap. Certains c'est un vu notifier une aide humaine ne sont toujours pas accompagnés d'autres pâtissent de nombre d'heures d'un compagnon inférieur à celui qui leur a été notifiée. D'autres encore voir leurs besoins non couverts par la quotité fixée cette carence de l'éducation nationale explique que certaines familles en arrive à rechercher par elles-mêmes ou par le biais d'associations des AESH dites privées un nouveau marché de l'accompagnement privé est en train de se développer.-- Même si là encore difficilement quantifiables mais cette évolution provoque une rupture d'égalité dans l'accompagnement du handicap et renforce les inégalités sociales. J'en viens en quelques mots à la situation des 67.000 assistants d'éducation. Également confrontés à des conditions d'emploi et de travail précaire. Au moment de la création de cette fonction, l'idée était d'en faire un tremplin pour d'éventuelles futures carrières dans l'Éducation nationale par le biais des concours de conseiller principal d'éducation ou de professeurs, force est cependant de constater qu'aujourd'hui le taux de réussite des à ED à ce concours est seulement de 15%. Et les étudiants représentent 30% des effectifs alors qu'ils étaient censés être majoritaire. Se pose dès lors la question du devenir professionnel des ED. Faut-il professionnaliser cette fonction pour permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à l'exercer d'en faire un véritable métier. Ou faut-il conserver là sa nature première et mieux garantir ses débouchés vers d'autres emplois. Ce débat de fond mériterait Madame la Ministre de mener un travail de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. En attendant, nous ne pouvons que constater et déplorer la grande précarité qui caractérisent aussi leurs conditions d'emploi et de travail des à Rémunération au niveau du SMIC grille indiciaire inexistante pluralité d'affectation, absence de formation et de perspectives professionnelles. Face à l'ampleur des enjeux que je viens de décrire pour partie commun à ces 2 catégories d'agents. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui se veut comme une première étape nécessairement modeste mais vers une amélioration de leurs conditions d'emploi et une reconnaissance du service qu'ils rendent à l'école inclusive. Son article 1er ouvrent la possibilité de recruter en CDI. Les AESH ayant exercé pendant 3 à 6 ans soit. Sein potentiellement à l'issue d'un seul CDD contre 2 actuellement exigé par la loi pour une école de la confiance. Alors que la très grande majorité des AESH enchaîne aujourd'hui les contrats courts synonyme d'instabilité et d'incertitude de précarité cette accélération de possibilité de céder nisation et gage de stabilité dans l'emploi de sécurisation du parcours professionnel et de reconnaissance professionnelle, elle est aussi une étape importante dans la professionnalisation du métier d'AESH et dans la construction de son attractivité. Notre commission a eu un débat sur la durée de la condition d'exercice exigé pour pouvoir prétendre à une CDI. Où placer le curseur à 3 ans comme l'a proposé l'Assemblée nationale, ce qui selon certains collègues la serait le temps d'évaluer les compétences professionnelles et permettrait de, de pas rigidifier le système pourquoi pas plus tôt dans la mesure où il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation qui permettrait aux. Ayant fait leurs preuves au bout d'un an de se projeter plus rapidement dans une carrière stable. Nous, nous sommes en tout cas tous retrouvés sur la nécessité de garantir l'effectivité de la formation initiale des AESH. Condition sine qua none à leur montée en compétences et professionnalisation. Notre commission a par ailleurs pleinement conscience que s'il a cédé. Ils assurent accéléré constitue une première avancée pour les AESH le chemin qu'il reste à parcourir pour améliorer leur statut. Et leurs conditions de travail est encore long. C'est pourquoi nous appelons collectivement le gouvernement a lancé sans plus tarder une réforme structurelle des conditions d'emploi des ASH dans le cadre de l'acte de de l'école inclusive nos estimant que plusieurs sujets relevant principalement du niveau réglementaire nécessite d'être travailler la quantité de travail dans le but de permettre aux AESH qui le souhait de travailler à temps complet, l'articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire. L'augmentation du niveau de rémunération qui passe impérativement par une revalorisation de la grille indiciaire l'application effective de la réglementation de l'éducation nationale en matière de remboursement des frais de transport, le renforcement de la formation et sa prise en charge financière. La révision de fonctionnement des pieds à la fin de remédier aux dérives constatées d'harmoniser les pratiques entre les territoires. J'en bien à l'article 2 de la proposition de loi, celui-ci ouvre aux à ED ayant exercé pendant 6 ans CDD le bénéfice du recrutement s'est dit en cas de poursuite de leur mission. Cette disposition votée par l'Assemblée nationale le 20 janvier dernier a entre-temps été satisfaites satisfaites par l'article 10 de la loi du 2 mars 2022, visant à combattre le harcèlement scolaire. Elle y a été introduite par le Sénat lors de l'examen du texte en première lecture à la suite de l'adoption de d'un amendement, présenté par notre collègue Toine. Pour éviter une redondance inutile. C'est vrai qu'il conviendrait de la supprimer mais sur ma proposition, la commission n'a pas souhaité le faire en effet les remontées de terrain font état de réticences de la porte de la part des rectorats au chef d'établissement a cédé Izé les a aidés. Après 6 ans de service sur la cible de 5000 CD nisation visé, seuls 1000 serait effective. Même si le décret d'application et publié le 9 août dernier, il ne il ne présente pas d'un d'ambiguïté une circulaire ministérielle serait peut-être nécessaire pour inciter les rectorats les chefs d'établissements à se saisir de cette disposition. Nous attendons que Madame donc madame la ministre, une réaffirmation du principe posé par la loi du 2 mars et un engagement de la part du gouvernement à être effective sur le terrain.-- Telle est le contenu des 2 articles qui composent cette proposition de loi que notre commission adopté à l'unanimité sans modification. J'émets le souhait que nos débats permet de quoi enfumer notre consensus autour de ce premier pas en faveur des AESH et qu'il ouvre aussi la voie à des avancées supplémentaires dans un avenir très proche. Je vous remercie. Merci. Dans Merci. Dans la suite de l'édition générale. La parole est à Madame, Samantha Cazebonne.--

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation sont des prêts, des pièces maîtresses des piliers de l'école inclusive. Cependant, ces pièces maîtresses sont aujourd'hui des pièces précaires dont la fragilité menace la solidité de cet édifice magnifique de cette fierté républicaine, l'école inclusive. J'entends par école inclusive. La mise en oeuvre de l'idée que le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap est un droit fondamental. Nous connaissons tous ici ces chiffres sans équivoque qui témoignent de la précarité de ces 2 métiers, plus de 80% des AESH exerce dans le cadre d'un CDD et seulement 2% d'entre eux dispose d'un emploi à temps complet. S'agissant de leur rémunération moyenne elle se situe autour de 850 euros Net par mois. Quant aux à ED. Ils sont aussi recruté par CDD sont rémunérés au niveau du SMIC et demeure une profession au devenir incertain. Ces chiffres sont d'autant plus regrettable que ces personnes qui sont pour la grande majorité des femmes aiment leur métier.-- Elles aiment accompagner quotidiennement les 400.000 élèves en situation de handicap que compte notre pays. À ce titre nombres d'AESH lorsqu'on les interroge sur leurs motivations, de leur métier évoque une forme de vocation. Le gouvernement a beaucoup investi en faveur de l'école inclusive depuis 5 ans puisque le budget dédié à cette dernière. A augmenté de 66% par rapport à 2017.-- Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a déjà amorcé la reconnaissance légitime des AESH. Ces derniers ont été reconnues comme des membres à part entière de l'équipe éducative et peuvent désormais participer aux réunions de suivi de la scolarisation des élèves en situation de handicap.-- En outre, c'est cette même loi qui a rendu possible leur CDI sation au bout de six ans de service et c'est encore elle qui a permis que des ED inscrits dans une formation préparant aux concours des métiers de l'enseignement et de l'éducation puisse exercer de véritables fonctions pédagogiques comme le font les personnels enseignants. Il y a enfin le budget présenté par le gouvernement pour l'année 2023 que nous venons de voter qui financent la création de quatre pardon de 4000 postes à ESH et une augmentation de 10% de leur rémunération. Le ministre a également annoncé que la prime Rep et Rep plus serait étendu pour les personnels exerçant en réseau d'éducation prioritaire dans le 1er et le second degré. Alors, en ouvrant la possibilité de recruter les AESH en CDI à l'issue. D'un seul CDD et en confirmant la possibilité de la CEDEAO sation des ALD cette proposition de loi, poursuit l'indispensable réforme de ces professions. Mais il faudra aller plus loin et engager une réflexion approfondie sur l'amélioration du statut et des conditions d'emploi des AESH. Je pense évidemment au sujet de la rémunération, mais aussi au renforcement de la formation à l'articulation entre le temps scolaire et le temps périscolaire et bien sûr à la CDU, nisation des AESH au bout d'un an pour toutes ces raisons, le groupe RDPI est très favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant madame Sabine Vanek pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure. Mes chers collègues. Je veux d'abord saluer la qualité du travail mené par notre rapporteure Marie-Pierre Monnier qui s'est trouvée confirmée par l'adoption de cette PPL à l'unanimité en commission jeudi dernier. La CDU nisation des accompagnants et accompagnante des élèves en situation de handicap à l'issue d'un seul CDD. Contre 2 aujourd'hui permise par l'article 1 de cette proposition de loi est évidemment indispensable, que les 132.000 AESH joue un rôle fondamental dans l'école inclusive pour assurer dans les meilleures conditions. La scolarisation des élèves en grande difficulté dans tous les établissements d'enseignement. Combien d'enfants seraient en échec total sans ce soutien de qualité est indispensable. Le CDI la norme dans notre pays et permet de se projeter dans l'avenir avec la possibilité de se loger d'emprunter. Rappelons qu'actuellement seulement 20% des AESH exerce dans le cadre d'un CDI c'est personnels ne bénéficient pas de la reconnaissance qu'il mérite. Leur rémunération est très faible en moyenne 850 euros par mois sous le seuil de pauvreté, avec des conditions de travail difficiles du temps incomplet subit des affectations de dernière minute parfois dans plusieurs écoles avec des frais de déplacement important peu pris en charge et pour certains le droit à la pause méridienne non respecté les AESH souffre également d'un manque de formation et il arrive que certains se forme sur leurs propres deniers, ou même que ce soit les parents qui finance les ces formations du fait de ses multiples difficultés on observe des phénomènes de démission de l'ordre de 10% et ce, au bout de deux 3 ans seulement. Le gouvernement ne prévoit pas assez de créations de postes d'AESH, 4000 seulement pour 2023 alors même que l'augmentation de prescription d'aide humaine pour 2020 et 2021 et de plus 12% sur la même période, le nombre d'AESH n'a augmenté que de 5%. Attention donc au recours à des AESH privés et donc à la rupture d'égalité. Il est primordial et urgent que le gouvernement, sorte de la précarité. Les 132.000 accompagnants essentiel dans la réussite de l'école inclusive et dont le nombre est amené à croître dans les années à venir. Ainsi, nous soutenons la demande de la rapporteur d'une réforme structurelle des conditions d'emploi des AESH dans le cas de l'acte de de l'école inclusive récemment annoncé par Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, les sénateurs socialistes avaient déposé de nombreux amendements au PLF pour aller au-delà de la CDU Lisa Sion et améliorer les conditions de vie et d'exercice des AESH 20 millions supplémentaires pour revaloriser les salaires alignement du montant des primes Rep et Rep plus des AESH pour les autres personnels de l'Éducation nationale, ouverture de 10.270 postes supplémentaires au lieu des 4000 prévues par le PLF. Nous attendions là un signal du ministre de l'Éducation nationale, mais nous ne sommes malheureusement heurté au véto tant de la majorité sénatoriale que du gouvernement. De la même manière. Monsieur le Ministre nous avait assuré que le gouvernement était favorable à une sédimentation au bout d'un an. Je m'étonne qu'aucune initiative de sa part en ce sens, ne se concrétise par le dépôt d'un amendement du gouvernement à la PPL dont nous d'hépato-. Cette proposition de loi entend aussi mettre l'accent sur la situation des 65.000 assistants d'éducation. ces délégations prévue par l'article 2 de cette de cette PPA permise grâce à un vote du Sénat. Depuis la loi visant à lutter contre le harcèlement scolaire et le décret du 9 août 2022. Il semble cependant que certains recteurs aux chefs d'établissement ils soient réticents et que seulement un 5ème des AE des susceptibles d'être cédées Izé les effectivement été d'où l'importance que le gouvernement réaffirme le principe et surtout l'obligation de la CDU des ED après 6 ans d'exercice. L'émission des ALD sont très polyvalente et leurs conditions de travail également difficile rémunération insuffisante différents lieux d'affectation, absence de formation. Le groupe du sénateur socialiste, écologiste et républicain soutient donc la demande de notre rapporteur, que le gouvernement engage une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, sur le devenir professionnel des assistants d'éducation. Nous avions déposé des amendements puis à lèvres 2023 visant à un alignement des primes. Plus et la mise au même niveau des rémunérations des ED de l'enseignement agricole et de l'enseignement général. Nous regrettons que ces amendements et eux aussi été rejeté en séance le 1er décembre dernier par la majorité sénatoriale avec l'accord du gouvernement. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne résoudra pas tout, et le chemin est encore long pour sortir ces personnels de la précarité, mais c'est un 1er pas. Le groupe des sénateurs socialiste, écologiste et républicain votera donc avec enthousiasme et lucidité cette PPL qui doit aussi être vu comme un appel à l'action du gouvernement, à qui nous demandons solennellement d'agir vite et fort sur ces enjeux primordiaux pour l'avenir de nos enfants et pour l'accession à l'emploi des personnels concernés dans des conditions dignes. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Nous voterons cette proposition de loi présentée par nos collègues socialistes que Marie-Pierre Monnier a pris l'initiative de mettre à l'ordre du jour, ici au Sénat, nous la voterons en regrettant que les députés de la majorité présidentielle, épaulés par ceux de LR. On est limité la portée. Nous la voterons en ayant à l'esprit tout le chemin qui reste à parcourir pour que les accompagnant de d'élèves en situation de handicap bénéficient d'une rémunération d'une formation et d'un statut digne afin que l'école inclusive deviennent une réalité pour tous. Trop d'enfants, trop de familles reste en effet encore sans solution longtemps c'est le manque de moyens accordés aux académies pour en recruter qui a été la principale cause aujourd'hui des postes créés ne sont pas pourvus, c'est le cas dans mon département de la Seine maritime comme dans bien d'autres les conditions statutaires, les conditions de travail et de rémunération offerte aux AESH en sont directement la cause. Or, je le rappelle l'inclusion et l'accompagnement des élèves en situation de handicap constitue une obligation de résultat pour l'État. Dans ce contexte, ouvrir la possibilité de recruter les AESH en CDI au bout d'un CDD de 3 ans plutôt que de six présente une avancée qu'il faut prendre. Mais soyons lucides sur le fait que ça n'est qu'une possibilité et que ça ne mettra pas fin réellement à la précarité. Quelle parce que ce sont vous le savez des femmes à plus de 90% les dès l'été dernier. Cette possibilité est ouverte pour le cru le recrutement des assistants d'éducation au bout de six ans de CDI et force est de constater qu'elle n'a pas tenu toutes ses promesses, puisque cela a été rappelé, seuls 1000 d'entre eux sur les 5000. Ont été réellement c'est déguisé et l'on peut craindre que les AESH connaissent malheureusement la même situation, tout en adoptant cette proposition de loi. Nous devons donc travailler à améliorer encore et très nettement leur sort c'est indispensable pour garantir l'accueil d'enfants et de jeunes en situation de handicap dans le milieu scolaire. Pouvons-nous accepter que la 2ème profession en termes d'effectifs au sein de l'Éducation nationale soit rémunéré sous le seuil de pauvreté après avoir été condamné à la suite d'une décision du Conseil d'État concernant les à ED. Le gouvernement a décidé d'octroyer des les primes. Plus aux AESH à compter du 1er janvier prochain mais elles sont inférieures à celles des autres personnels de l'éducation et la rémunération des AESH restera plus faible que le seuil de pauvreté, y compris après l'augmentation de 10% qui leur est promise à la rentrée 2023. La mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localiser ces fameux pial, répondant à une logique de mutualisation des moyens entre établissements est censée accroître leur temps de travail essentiellement des temps de travail partiel subi n'a pas à améliorer la situation, au contraire. Quant à leur formation, elle reste elle aussi à développer. Si l'on veut professionnaliser les AESH et leur donner toutes les compétences compte toutes les compétences nécessaires à l'accueil d'enfants aux situations et aux besoins très divers à l'aube de l'acte de de l'école inclusive annoncé par le ministre de l'Éducation nationale et alors que se pose la question de l'accompagnement des enfants en situation de handicap en classe mais également durant toutes leurs activités d'enfants. Il nous semble urgent de mettre sur la table l'intégration des AESH à la fonction publique ce statut qu'il convient de moderniser plutôt que de le détériorer permet en effet des passerelles entre collectivités et État il pourrait être un creusés à même de répondre aux besoins que nous identifions et de créer le cadre national nécessaire face aux disparités de situation que nous connaissons d'un département à l'autre. Il permettrait aussi de mieux intégrer les AESH aux équipes éducatives dont elles font, à nos yeux pleinement partie pour accompagner, enfants et jeunes. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant à madame Annick Billon pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure chers Marie-Pierre. Monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. Le texte que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de lutter contre la précarité de 2 catégories de personnels de l'éducation nationale les accompagnants d'élèves en situation de handicap et les assistants d'éducation à la rentrée dernière. L'éducation nationale recensait 132.000 AESH dont 93% de femmes. Les AESH et les à ED non pas tout à fait les mêmes missions mais les uns comme les autres sont confrontés à des conditions de travail extrêmement précaires parmi les causes de cette précarité, je citerai les conditions de recrutement 80% sont recrutés en CDD. Le temps partiel, seuls 2% des AESH dispose d'un emploi à temps plein pour la majorité ce temps partiel est un temps partiel subi, obligeant certains à cumuler plusieurs emplois. La rémunération n'est en moyenne que de 850 euros mensuels la formation actuellement 60 heures de formation sont prévues par les textes 16h qui peuvent se réaliser à la fois en présentiel ou en à distance. À priori, s'apparente plutôt à une boîte à outils. Les formations initiales comme continues font donc défaut et cela peut contraindre les avais sage à s'auto former dans certains cas même d'ailleurs ce sont les familles des enfants accompagnés qui paye une formation. Ceci n'est évidemment pas acceptable et c'est pourquoi j'ai déposé 2 amendements concernant la formation. Ces amendements sont avant tout des amendements d'appel qui doivent permettre d'entamer un échange avec vous madame la ministre, la discussion que nous avons eu lors du projet de loi de finances et plus particulièrement lors de l'examen de la mission enseignement scolaire ne ne nous ont pas satisfaits et c'est un faible mot affectation dans différents établissements du territoire du pial de rattachement accompagnement simultanée de plusieurs enfants présentant souvent des pathologies différentes. Frais de déplacement qui ne sont pas pris en charge ou même parfois accomplissement de tâches qui ne font pas partie d'émission de ces métiers. Lors des différentes auditions auxquelles j'ai pu assister avec madame la rapporteure. Le constat a été souvent le même, des conditions de travail de plus en plus dégradé viennent s'ajouter à la précarité de l'emploi et celle-ci mène de plus en plus à des arrêts maladie à répétition ou même à des démissions. En 10 ans le nombre d'élèves en situation de handicap, scolarisés en classe ordinaire a connu une augmentation de 60% dans le primaire et de 150% dans le secondaire. Pour faire face à à cette hausse. 4000 AESH supplémentaires et des efforts budgétaires substantielles oui ont été réalisées. Malgré cette hausse bienvenue, force est de constater que de nombreux élèves en situation de handicap ne sont pas accompagnés ou mal accompagné.

Pour les, des, les conditions de travail sont tout aussi précaire. Si cette fonction dont le statut n'a pas évolué depuis 2003. Il a été pensé d'ailleurs à ses débuts pour les étudiants, l'âge moyen des assistants d'éducation est aujourd'hui de 30 ans donc, nombreux sont ceux qui ont à leur charge une famille. Ces dernières années, beaucoup d'entre eux ont démontré une volonté de se professionnaliser et de sécurité leur de sécuriser pardon leur parcours sur le long terme. À ce stade il n'ont pourtant pas la possibilité d'accéder à un CDI. Ils sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de nos établissements et à la lutte contre le harcèlement scolaire par exemple, mes chers collègues. Ce texte marque une étape dans la lutte contre la précarité des métiers à ESH et à ED. Mais ce n'est qu'une première étape. Trop de dispositions relèvent du réglementaire et ne nous permettent pas d'activer véritablement les leviers nécessaires pour faire évoluer leur situation. L'éducation nationale doit train entamé un travail de fond pour permettre une évolution plus que nécessaire des conditions de travail de ses chevilles ouvrières de l'école inclusive.

avant de conclure, je voudrais saluer le travail précis et de qualité de notre rapporteur Marie- Pierre Monnier sur ce texte qui je l'espère permettra d'ouvrir une vraie réflexion sur ses métiers essentiels. Enfin la création d'une mission d'information sur les modalités de financement, et la mise à disposition d'AESH sur le temps de la pause méridienne et d'accueil périscolaire. Autre point de difficulté important apportera des réponses peut être complémentaire à cette reconnaissance. Nous serons très attentifs à ces ce conclusion mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera avec enthousiasme pour ce texte, madame la rapporteure en espérant qu'il sera le point de départ d'une vraie évolution pour les AESH et les Alder je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, monsieur le président de la commission. Mes chers collègues. En politique la vertu et de mettre en cohérence, son éthique de conviction et avec son éthique de responsabilité. Et en soutenant cette proposition de loi conforme sans amendement nous sacrifions un peu à notre esprit de responsabilité. Mais c'est pour faire progresser la condition des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et puisqu'une unanimité de sagesse choisi la voie du petit pas du compromis plutôt que la quête du grand soir. Eh bien vous comprendrez que le groupe RDSE se joindra à la modération sénatoriale légendaire. Puisque nous ne reviendrons pas sur la forme. Cela me permet d'exprimer quelques réflexions sur le fond. L'intégration scolaire des enfants porteurs de handicap est une belle et noble idée. L'accompagnement de ses enfants par des AESH Elisa ED est également une belle intention. Cette école inclusive permet à des enfants de progresser de s'épanouir et à d'autres de s'enrichir en côtoyant les différences et en les intégrant. Elle permet également. Dans certains cas, d'offrir des activités enrichissantes à temps partiel parfois à temps complet à des échos à des accompagnants qui peuvent ainsi exercer une activité qu'il n'avait pas forcément envisagé et percevoir un complément de revenu familial utile et qui a du sens. Mais je sais que tout n'est pas aussi toujours idyllique et que la précarité de ces emplois et les lourdeurs des tâches peuvent mettre en souffrance celles et ceux qui les subissent. Car le balancier de l'école inclusive et peut être remonter trop haut. Certains handicaps sont trop lourds pour l'inclusion scolaire même accompagner au mieux. Ils mettent en souffrance l'enfant l'accompagnant les autres enfants de la classe et les enseignants. Ce remarquable dispositif d'inclusion ne convient pas à tous les handicaps et les associations de familles d'enfants porteurs de handicap nous alerte Madame la Ministre sur le besoin de places supplémentaires en IME qui répond davantage aux besoins de handicaps plus lourds. Avec une bonne orientation en IME avec des places d'accueil disponibles. Et en inclusion à l'école pour les handicaps compatible, nous répondrons à cette souffrance induite et nous rendrons humainement supportable la tâche des accompagnements, des Enfin. J'en profite pour plaider pour que les départements avec leur MDPH prenne la main sur les AESH et à ED pour une gestion cohérente et proximité du handicap par leurs services médicaux sur Sio qui assure déjà le dépistage et l'accompagnement social des familles. C'est un des domaines dont il faut délester l'éducation nationale qui doit être plus ouverte aux collaborations avec les collectivités locales en fonction de leurs compétences. C'est un autre chantier mais j'en profite pour le rappeler.-- Je vous remercie. La parole est maintenant monsieur Philippe mouiller pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame le Ministre.-- C'est le prendre la commission madame la rapporteure, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation. Il s'agisse déjà été dit de permettre aux et messages d'être recruté en CDI au terme de leur 1er CDD de 3 ans et aux assistants d'éducation ayant exercé pendant 6 ans leur activité, d'être recruté dans le cadre d'un CDI. En 2022 au comptait plus de 135.000 ASH et environ 65.000 à ED. La même année, le nombre d'enfants en situation d'handicap accueilli en milieu ordinaire était de plus de 400.000. Il faut souligner l'effort financier et l'effort de recrutement de l'Éducation nationale. Les moyens sont conséquents. Mais les, j'ai dit il existe un très fort décalage entre l'objectif annoncé par le gouvernement sur l'inclusion scolaire et les résultats sur le terrain. Oui, un trop grand décalage entre l'augmentation des moyens humains et financiers en faveur de l'accompagnement des élèves et le nombre croissant d'enfants dont les besoins ne sont pas ou mal couverts. La promesse faite aux familles concernées par le handicap ne peuvent être tenus dans ces conditions.-- Partout dans le territoire. Nous avons heureusement des bonnes réalisations.-- Des situation satisfaisante mais également de trop nombreux jeunes qui ne peuvent bénéficier de l'accompagnement humain dont ils ont besoin. Faute de budget ou du personnel disponible. De plus, les conditions de travail et le métier d'AESH reste précaire et trop peu attractif. Par manque d'heures de travail de 24h par semaine en général les niveaux de rémunération sont très faibles, environ 850 euros Net par mois, même si des évolutions soient attendues dans les mois qui viennent. Les AESH ne bénéficient pas toujours de formation adaptée et sont souvent mal intégrés à la communauté éducative. À cela se rajoutent des problèmes de dialogue. Point essentiel problème du dialogue entre l'éducation nationale, le médico-social et les MDPH entraînant des situations difficiles pour les accompagnants et les enfants suivis. Dans mon département, j'ai eu connaissance de nombreux exemples des messages qui découvrent une semaine avant la rentrée scolaire le ou les établissements dans lesquels ils sont affectés. Le nom de l'enfant en situation de handicap et surtout la nature du handicap de l'enfant.-- Dans ce contexte, comment une personne, quelle que soit sa bonne volonté peut-elle accompagner de façon satisfaisante. Un jeune autiste. Puis l'année suivante un enfant concerné par Nice sans formation et sans préparation.-- En complément, la loi pour une école de la confiance a permis la mise en place des pial. Cette nouvelle forme d'organisation du travail des AESH devait permettre de mieux répartir et coordonner leurs interventions en fonction des besoins et des emplois du temps des élèves concernés. Mais la réalité est tout autre. Car dans beaucoup département très souvent c'est pour plutôt la gestion de la pénurie de moyens qui est organisée par les Aujourd'hui, quel bilan positif. Pouvez-vous établir de la réforme qui était installé les pièces sur tout le territoire d'une bonne idée d'un principe général de coordination. Le manque de moyens entraîne une autre mission des pial. Malgré la bonne volonté des pouvoirs publics. Le système n'est pas pleinement satisfaisant. Entraînant un manque d'attractivité du métier d'AESH a été dit, des situations sociales difficiles et un accompagnement des enfants en situation de handicap imparfait. Une véritable réforme s'impose. Avec comme objectif principal de mettre le parcours de l'enfant au centre du dispositif. Et on ne peut résumer les choses simplement en disant que lorsque nous n'avons pas surnomme moyens les établissements, les instituts de la bonne réponse. Il faut vraiment avoir analyse globale du parcours de vie de l'enfant.-- On peut notamment se poser la question aujourd'hui clairement. Est-ce que l'éducation nationale est aujourd'hui le meilleur gestionnaire de l'inclusion scolaire ou ne faut-il pas s'appuyer davantage sur le médico-social.-- Comment améliorer le dialogue entre ces 2 mondes qui ont tout de même en commun, l'intérêt de l'enfant accompagné. Comment améliorer l'organisation sur le terrain et mettre en place un statut professionnel satisfaisant pour les AESH finalement comment rendre ce métier attractif. De nombreuses questions qui restent aujourd'hui incomplète dans leur réponse. Concernant la proposition de loi que nous examinons le groupe politique s'est beaucoup interrogé sur le vote exprimé car voté favorablement risquerait peut-être d'inscrire dans le marbre et valider la situation précaire de ces agents de l'Éducation nationale. Cela risque d'être un moyen de pérenniser un système qui aujourd'hui est défaillant.-- Malgré cela et pour envoyer un signe positif aux agents dont nous reconnaissons la qualité du travail. Nous voterons cette proposition de loi, tout en exprimant un voeu fondamental pour la mise en place d'une véritable réforme de l'inclusion scolaire c'est un objectif que nous avons en commun les moyens sont sur la table les résultats attendus aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. Je vous remercie.

Madame la présidente, madame la ministre madame le rapporteur. Mes chers collègues. L'école inclusive vise à assurer de scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée lycée partout et pour tous. Cette belle ambition fait partie des priorités annoncées par le président de la République pour le mandat en cours. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont les pierres angulaires de la bonne intégration des élèves porteurs de handicap raison d'être de l'école inclusive. ces accompagnant on vit aujourd'hui dans une situation de grande précarité ce ça n'est pas acceptable. En moyenne vous avez perçoivent un salaire moyen de 850 euros par mois en deçà du seuil de pauvreté. Cette rémunération est évidemment insuffisante pour vivre décemment et les obligent parfois accumuler d'autres emplois à temps partiel. Le contexte inflationniste accentuent la gravité de la situation et nous engage à agir. Le 22 janvier 2022. La proposition de loi pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier 1er décembre la commission de la culture, d'éducation et de la communication a également adopté le texte à l'unanimité. Je salue l'approche collégiale et transpartisane dont le Parlement a fait preuve. Le premier article ouvrent la possibilité de recruter en contrat à durée indéterminée. Les AESH après 3 ans d'exercice, c'est-à-dire à l'issue d'un seul contrat à durée déterminée. Par ce texte nous déposons une première Pierre pour l'amélioration des conditions de travail des accompagnants. Cette avancée est modeste, certes, mais elle va dans le bon sens. Une contribution du Sénat dans la loi visant à lutter contre le harcèlement scolaire a déjà permis de ces. Les assistants d'éducation à la suite de de CDD. Pourtant certains chefs d'établissement refuse encore de mettre en pratique cette avancée sociale comme le prouvent les remontées de terrain. Le vote de cette proposition de loi réaffirmera. Je l'espère. Ce dispositif pour endiguer la précarité dont souffrent également les assistants d'éducation. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une revalorisation salariale mais aussi la création de 4000 nouveaux postes USH à la rentrée scolaire 2023. L'augmentation des effectifs est une bonne chose, tant les besoins sont en augmentation constante. À ce jour, 44% des élèves en situation de handicap ne bénéficient pas d'un accompagnement humain pourtant essentiel pour les accompagner dans les pratiques quotidiennes le travail scolaire et les activités relationnelles. Derrière ce taux abstraits. Ce sont des milliers de jeunes dépourvus de la présence d'un accompagnant à leurs côtés. Pour autant, ces mesures de peuvent nous satisfaire tant les enjeux en matière d'amélioration des conditions de travail de développement du recours au temps plein et de rémunération sont immenses. La grande disparité des situations observées en fonction des territoires, nous interpelle et souligne l'urgence de l'harmonisation des pratiques enfin. La qualité de l'accès à l'information est essentiel, tant pour les AESH eux-mêmes que pour les jeunes en situation de handicap nécessitant un accompagnement spécifique. Notre groupe les indépendants République et Territoires votera favorablement ce texte et appelle à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Cette proposition doit marquer le lancement d'un débat d'ampleur sur l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école. À ce titre, nous serons attentifs aux travaux prévus en amont de la conférence nationale sur le handicap annoncé au printemps 2023. Je vous remercie.

Madame la présidente madame la rapporteure Madame la Ministre, mes chers collègues. La situation des accompagnants d'élèves en situation de handicap dans notre pays est un scandale absolu. Absolu. Plus de 130.000 femmes, la profession est. Féminine à 93% exercent une mission indispensable auprès des enfants en situation de handicap sans leur travail, ces élèves ne pourraient pas suivre une scolarité comme les autres élèves. On parle donc ici de l'essentiel du non négociable de quelque chose de vital dans notre pacte républicain, oeuvrant pour une politique indispensable pour une école ouverte à toutes et tous. Elles sont méprisés par l'État employeur comme bon nombre de travailleuses et de travailleurs essentiels ces ESH exerce dans des conditions indignes. Leur salaire moyen autour de 800 850 euros par mois bien en dessous de tous les seuils de pauvreté relative ou absolue, cette faible rémunération est en grande partie due à une incapacité systémique de ses personnels à travailler à temps plein. L'organisation de travail et notamment en raison de trop grands pial qui les forces et mobilité importante ne permet pas d'atteindre les 35 heures en moyenne, les AESH passe 24h par semaine auprès de leurs élèves. Le reste du temps elle le passe sur les routes. Seulement 2% des messages sont à temps complet de Leur statut ou plutôt l'absence de statuts est devenue un enjeu de premier ordre. 80% des AESH accumulent les CDD, ce qui les plonge dans une grande précarité subie. Ajoutons à cela une faible formation des incertitudes bureaucratique sur pour savoir qui de l'État ou des collectivités doivent prendre en charge les temps périscolaires souvent en une exclusion de l'équipe pédagogique voilà réuni toutes les conditions pour saper pour décourager à petit feu une profession toute entière. Ce n'est pas du catastrophisme. Le système actuel, ils avaient sache nous monte des premiers signes d'effondrement. Il y a 2 fois plus d'enfants en situation de handicap ayant besoin d'une aide humaine dans notre pays que d'AESH ses enfants se retrouvent bien souvent sans solution à tel point que les familles qui peut ont désormais recours à des AESH privés pour pallier leur manque une rupture d'égalité insupportable symptôme de l'urgence de la situation. Vient ensuite. La question des assistants d'éducation les AED. Si leur situation est moins critique que celle des AESH. Elle doit aussi nous alerter cette profession était pensé au départ comme une première immersion dans la communauté éducative pour des jeunes qui aurait vocation à se présenter ensuite aux concours de CPO de professeurs, aujourd'hui seuls 15% des. S'engage dans cette voie et moins d'un tiers sont des étudiants. Nous avons donc des gens qui pour qui être à ED devient peu à peu le métier alors que la profession est tout aussi précaire que celle des AESH. Voilà comment on traite aujourd'hui, des personnels de l'Éducation nationale, dès lors que faire sur proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'attaque un premier problème le statut certes il il s'y attaque à la marge mais ce n'est pas la faute des auteurs du texte. Revenons en décembre 2021, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale dépose un texte prévoyant le recrutement des AESH en CDI avec un coffre coefficient de pondération de 1,2 pour reconnaître le temps de préparation pour les AE dès l'été prévu une possibilité de recrutement en CDI avec l'obligation de les recruter au bout de six ans. Six qu'un taux d'encadrement minimal pour les AESH. Il est enfin prévu l'accès aux primes Rep et Rep le texte qui nous arrive aujourd'hui a été largement vidée de sa substance. Après son passage à l'Assemblée. La faute à une majorité présidentielle bien majoritaire à l'époque et qui trouvait que le texte allait trop loin. Le texte d'aujourd'hui prévoit seulement que les avait sache. Puisse être recrutés en CDI dès la fin de leur 1er contrat de 3 ans et que les a aidés puisse être recrutés en CDI au bout de six ans. Toutes les dispositions relatives à l'encadrement et à la pondération sont supprimés. Comble d'ironie certains concernant les l'article ne change strictement rien à la législation actuelle on en vient simplement espérer une confirmation du droit, a-t-elle par la ministre en séance. Drôle de façon de légiférer ou plutôt de ne pas légiférer alors oui le groupe écologiste votera ce texte car nous prenons chaque pas en avant chaque avancée si infime soit-elle pour améliorer le sort des personnels de éducation mais nous regrettons très vivement les manoeuvres politiques qui ont qui ont été menées pour vider ce texte. Je vous remercie.

Madame la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues.-- Nous vivons dans un pays, la France qui est souvent tenté par la division est accoutumé à à la polémique. Il y a pourtant un sujet qui fait consensus. Le droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants et cela quel que soit leur handicap.-- Depuis la loi de 2005 sous l'impulsion de Jacques Chirac. La prise en compte du handicap sa prise en charge et son accompagnement est désormais une priorité nationale et un défi pour chacun et chacune d'entre nous. Depuis 2013, le principe de l'inclusion scolaire pour tous les enfants sans aucune distinction figure à l'article 1er du code de l'éducation.-- D'énormes progrès ont été faits depuis ces dates. Pourtant, nous sommes encore. Loin d'être arrivé au bout du chemin.-- Cette proposition de loi. Déposée à l'initiative du groupe socialiste et visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation a été adopté la semaine dernière à l'unanimité par la commission de la culture de l'éducation et de la communication sans aucune modification.-- Il ne constituent probablement pas une grande avancée. Mais il est un 1er pas. Un 1er pas fait dans la bonne direction. Il est aussi un message positif envoyé en direction des AESH qui travaillent dans des conditions difficiles. À l'accompagnement des enfants en situation de Audi du handicap au quotidien.-- C'est pourquoi les élus du groupe les républicains et apparentés le votera comme je l'espère l'ensemble des membres de notre assemblée. Nous souhaitons aussi que ce texte puisse être voté conforme. Afin qu'ils puissent rapidement être mise en oeuvre car la tentation que nous avons tous eu à un moment ou à un autre. De pouvoir l'amender. Le condamnerait en fait à se perdre dans une nouvelle navette parlementaire, à l'issue lointaine et incertaine.-- Je voudrais. Remercier particulièrement. Notre collègue Marie-Pierre Monnier.-- Rapporteur de ce texte pour le travail et les échanges et les échanges que nous avons eu lors des auditions auxquelles j'ai plaisir à participer qui nous ont permis d'approfondir le sujet bien au-delà du texte qui nous rassemble aujourd'hui. J'aurais d'ailleurs l'honneur dans les prochaines semaines de pouvoir approfondir ce travail au sein d'une mission spécifique que je mènerai au nom de la commission de la culture et l'éducation et je remercie donc au passage le président Laurent Lafon et mon collègue Max Brisson pour leur confiance.-- Notre pays compte aujourd'hui 430.000 enfants scolarisés reconnues en situation de handicap. Ce chiffre a quadruplé durant les 20 dernières années. Ils représentent environ trois et demi pour 100 de l'ensemble des effectifs scolaires, soit en moyenne un enfant par classe.-- Le ministère de l'Éducation nationale emploie 130.000 AESH faisant de après les enseignants, le 2ème métier le plus important de ce ministère, j'utilise le mot métier à dessein. Car il est justement plus que venu le temps de faire de ces missions d'AESH un véritable métier.-- Il est temps de passer d'une logique purement quantitative, à une approche plus qualitative. Il est temps Madame la Ministre de mettre enfin de la justice, de l'ordre et de l'organisation dans l'accompagnement des enfants et des adolescents concernés. N'oublions pas qu'au coeur de ce débat. L'objectif poursuivi et la réussite de la scolarisation des enfants en situation de handicap et pour cela les aides humaines sont essentielles et nécessaires. Cependant, elle ne doivent pas être l'unique réponse pour une école inclusive d'autres solutions et moyens supplémentaires sont nécessaires pour que l'environnement pédagogique permettent cette inclusion scolaire en adaptant le matériel pédagogique et les espaces d'enseignement par exemple mais aussi en adaptant la pédagogie ou encore en améliorant la formation des enseignants. Le lien avec le secteur médico-social, mon collègue Philippe mouiller la rappeler tout à l'heure est aussi incontournable et constitue probablement une condition sine qua non de la réussite de cet accompagnement dans les années futures. Concernant l'accompagnement humain il n'est pas concevable de poursuivre dans la voie actuelle avec un système complexe flou sans véritable cadre national pour le recrutement des personnels ou l'affectation auprès des enfants et avec trop peu de différenciation pour adapter l'accompagnement collectif ou individualisé nécessaires au suivi de chaque enfant. Un système qui s'appuie enfin sur des agents désormais très nombreux mais qui sont insuffisamment insuffisamment accompagné pour être professionnalisées mieux formés et qui se retrouve le plus souvent enfermés dans une énorme proportion dans une situation de précarité indignes de l'État.-- L'accélération de la civilisation permettra, donner un peu plus de stabilité et un début de reconnaissance. Il reste encore beaucoup d'autres questions particulièrement depuis que le Conseil d'État à la demande du ministère de l'Éducation nationale, rappelons-le à scinder l'organisation du temps scolaire et du temps périscolaire entre l'État et les collectivités. Revenant sur cette règle qui semblait acquise jusqu'ici que tout ceux qui concourait à l'inclusion scolaire était de la compote de la, de la compétence de l'État. Cette décision est lourde de conséquences pour les collectivités comme pour les AESH. Et vu que je suis en retard, je vais accélérer. Et j'ai, j'ai appris ce matin fort opportunément par le le ministre de l'Éducation nationale qu'une circulaire. Allait dans les tout prochains jours être prises pour permettre justement cette prise en charge cet employeur unique qui permettra à ces à attaques d'avoir un employeur unique d'avoir un contrat unique et et de régler un certain nombre de problèmes, c'est une attente forte de la part des collectivités. C'est une avancée sur laquelle nous. Nous nous étions nombreux à l'attendre toutefois et il est maintenant nécessaire de mettre sur le, le métier. Le chantier de la réforme et de la professionnalisation de ces ESH, je vous remercie. Merci la discussion générale est Close et nous passons maintenant la discussion du texte de la commission à l'article 1er, une demande de parole de madame Françoise Gatel.-- Dames. La présidente Madame la Ministre je voudrais d'abord saluer cette initiative sur un sujet. Majeur et essentiel, et je voulais remercier le président la font et Cédric Vial et Max Brisson pour la mission qui lance, Au nom de la réflexion que nous avons conduites dans DS. Sur l'efficacité de l'action publique et le sujet dont nous parlons relève aussi d'une chaîne de décision ou de mise en oeuvre qui n'est pas opérante aujourd'hui. Je rappelle que la décision d'accompagnement d'un enfant handicapé relève de la MDPH, qui signifie cela à l'éducation nationale qui elle sollicite des crédits auprès de l'ARS à tout moment de l'année et que les communes elles-mêmes se retrouve dans un vide sidéral parce qu'elles n'ont pas les ressources pour des raisons diverses et variées, donc je pense qu'il faut améliorer l'organisation. Du système et qu'il faut effectivement professionnaliser ces curés sécurisé pardon ce personnel remarquable et les enseignants et rendent c'est le. Cette profession plus attractive. Vos mesures le permettent. Mais je pense et j'aimerais que l'on poursuive la réflexion sur un transfert sous réserve naturellement du volontariat des départements de petite de l'expérimentation et de transferts de moyens de la création dans des, dans les départements de services mutualisés. Qui pourraient être mises à disposition et de l'éducation nationale et des communes parce que chacun de nous connaît la situation de communes qui habitent très loin d'une ville et qui doivent trouver pour l'heure du déjeuner, c'est-à-dire une heure et demie du personnel pour accompagner les enfants, cela relève même pas du miracle, c'est juste impossible donc merci, Monsieur le président. De cette réflexion que nous nous poursuivons notre code que mais nous le ferons en échange. Dans le cas du groupe de travail que le président Larché a lancé, merci beaucoup.-- Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Je salue également cette proposition de loi mais je voudrais faire un pas de côté. On constate depuis des années une explosion des dossiers déposés sur les bureaux des MDPH, on constate une explosion des troubles du comportement, des troubles des apprentissages. Les études s'empilent on connaît une partie des responsabilités, elles sont. Mais il y en a 2 qui ressortent. La première concerne le temps passé devant les écrans de la 2ème ce sont les perturbateurs endocriniens effectivement cette explosion. Si on ne la traite pas. On s'en sortira pas. Alors bien entendu, aujourd'hui on est en train de chercher des des Budgets recherche déséquilibre parce que effectivement tout cela a un coût. Moi je propose que, hé bien les responsables de ces perturbations soient également les payeurs et qu'on instaure des taxes sur ces choses qui viennent altérer la santé mentale de nos enfants. Aujourd'hui on est dans une situation où il y a une maltraitance une maltraitance. Palpable auprès des AESH des AUD des enfants et des parents, il faut se sortir de là et je pense qu'il va falloir mettre des Budgets conséquents et aussi traiter le problème à la source. Juste une petite intervention rapide. Suite à l'échange de notre collègue. Je pas sur la motivation simplement un point de détail. Si dans nos débats au niveau du sénat on considère que le handicap étant une coïncidence, c'est une maladie. Alors dans ce cas il faut tout revoir, il faut tout refaire. Voilà je voulais juste préciser, à un moment donné il peut avoir des incidences liées à la maladie mais le dit qu'avant tout c'est des situations et l'inclusion c'est l'intégration cette différence et c'est pas une incidence de maladie.-- Très bien. Nous sommes saisis à l'article 1er d'un amendement de Mannheim Billon.-- Merci madame la présidente. Donc c'est un amendement d'appel et lorsque je je l'ai évoqué, et ça a été évoqué par d'autres interventions non dans la discussion générale. Il vise à insister sur la formation qu'elle soit initiale et continue, on l'a vu au cours de nos auditions et la rapporteure la constater, parce qu'il y a des départements exemplaire madame la rapporteure. Mais il y a des départements où cette formation mise mise finalement en application à géométrie extrêmement variable. Donc oui la CDI sation est quelque chose qui est important dans un pas pour la reconnaissance de ces métiers et on l'a tous disent tous ces sur mais on ne pourra pas imaginer dans le long terme. Une CDI sation sans une formation solide obligatoire et efficace, qu'elle soit initiale et continue, donc c'est l'objectif de cet amendement parce que CDI sation ne fera pas tout pour la reconnaissance d'un métier essentiel c'était c'est le sens de cet amendement et j'aimerais. Puisque nous en avons discuté en commission. Monsieur le président de la commission j'aimerais véritablement je connais la position de la rapporteure. Par rapport à l'amendement, nous partageons le constat. nous sommes tous d'accord pour faire ce pas. Un 1er pas vers les AESH. Mais ce pas n'est pas suffisant donc Madame la Ministre j'attends de savoir qu'est ce que va être par exemple l'acte de qu'est-ce que vous allez proposer parce que comme le disait Céline Brulin, au moment de la discussion générale, tous les amendements qui portaient des améliorations pour les AESH au cours du PLF ont été balayés Nat revers de ma mère. Oui c'est vrai que à partir du moment où on en CDI, on a besoin d'une formation et c'est vrai que dans les auditions qu'on a vu, on s'est rendu compte qu'en effet, d'un département à l'autre, il n'y avait pas les mêmes. Formations qui a été mise en place. Néanmoins, c'est dans la loi, la loi elle est déjà écrite. C'est le bénéfice d'actions de formation continue est prévue dans l'article L 917 tirer 1 du code de l'éducation et c'est pas Pas un manque au niveau législatif, mais plutôt c'est son application sur le terrain qui ne va pas et donc c'est au Service académique à qui revient de veiller à l'effectivité de l'accès des AESH, la formation continue en particulier aux Module de formation spécifique à l'accompagnement des élèves en situation de handicap qui sont prévus dans les plans académiques et départementaux de de formation. Donc c'est vrai que cet amendement. Madame la ministre et pour nous enfin et pour les auteurs en tout cas une alerte qui est qui est posée pour sur la nécessité de garantir vraiment l'efficacité. Néanmoins, chers collègues, je vous demanderai le retrait de cet amendement. Sinon ça serait un avis défavorable. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Je voudrais d'abord j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer à la fin de la discussion générale sous d'abord vous remercier. Pour la richesse de ces débats. Pour en fait avoir constaté. Que nous sommes tous unanimes sur le fait que, d'abord premièrement que les avais sage sont des personnels précieux. Deuxièmement qu'il nous faut conforter leur statut renforcer l'attractivité des métiers et faire en sorte. De de de pouvoir compter sur ses personnels précieux. Avec plus de sérénité pour ces personnels qui sont eux importants pour. L'accès à l'autonomie de nos, de nos enfants. En situation de handicap. Alors vos débats ont largement dépassé les AESH. Et vous avez parlé alors je veux je veux le dire très rapidement je je vous prie de de m'excuser. Madame la présidente. Mais je, je profite de l'occasion. Vous avez parlé. De la prochaine conférence nationale du handicap de sa préparation il y a effectivement des groupes de travail qui sont à l'oeuvre au ministère de l'Éducation nationale pour le sujet de l'école inclusive et de ce 2ème acte de l'école inclusive et il y a des représentants des parlementaires. Enfin il y a des parlementaires présents dans les groupes de travail donc j'encourage voilà ces parlementaires aussi. Ah vous faire passer l'information. De de ces travaux. Sachez que nous sommes très motivés pour poursuivre pour organiser pour aussi rapprocher le médico-social de l'éducation nationale qui est un un pan important et qui nous permettra d'avancer, je pense. Dans le. L'organisation de cette école inclusive. Donc nous avons il y a 2 grands pas qui ont été faits et je crois que l'on peut s'être heureux. De constater aujourd'hui qu'il y a plus de, enfin il y a 2 fois plus de fois et demie plus d'enfants qui rentrent dans le secondaire comme primaire aujourd'hui, ce qui montre que les enfants en fait suivent. L'école primaire et ensuite il passe au collège et ensuite il passe au lycée avec une augmentation importante de nombres d'enfants qui passent des brevet des collèges et qui passe des baccalauréats des enfants en situation de handicap. Donc je pense que l'école inclusive. Même si elle a beaucoup d'imperfections encore aujourd'hui c'est quand même une réussite et il faut que nous poursuivions inlassablement avec une organisation différente pour qu'elle soit encore meilleure et encore plus inclusive pour tous les enfants. Pour répondre à la question concernant la formation, la formation est essentiel, essentiel pour les AESH, on en a parlé aussi pour les enseignants et je crois pour tous les personnels qui sont dans les établissements, y compris pour les personnels municipaux dans les écoles pour les personnels. Départementaux dans les collèges et pour les personnels régionaux dans les lycées. Afin de sensibiliser chacun au handicap et à la façon. De. Bien de se comporter de prendre en charge certaines situations qui peuvent se produire à tout moment dans les établissements en tout cas. Les AESH ont besoin bien sûr de formation. Il y a 60 heures de formation qui sont dédiés à la formation de prise de poste et ensuite bien entendu il y a la formation continue. La formation continue qui êtes inscrites de vous l'avez dit dans le le code, vous l'avez dit madame la rapporteure. Et donc. L'accès à cette formation continue. Elle doit être renforcée. Et ces formations ne vont être renforcées avec notamment des formations communes aux enseignants et aux AESH afin de de de donc renforcer leur intégration au sein des équipes éducatives. vous avez raison, il s'agit de de de renforcer ceux là tant au niveau initiale que continue mais il faut que s'assurer de la, de l'accès effectif des agents à ces formations et au bon moment. je crois que ça c'est absolument essentiel et l'éducation nationale bien sûr, travail, travail sur ce sur ce sur ce sujet donc on partage vos. Vos objectifs mais les mesures en place permettent d'ores et déjà. De préparer les ESH à leur entrée dans le métier et d'autre part de développer leurs compétences. Par la formation continue, inscrite dans le code de l'éducation. Donc comme Madame la rapporteure. Je vous remercie. Si vous acceptez de le retrait de votre amendement sinon j'aurais un avis défavorable, parce que j'estime que. Dans les choses sont réalisés.-- Merci madame la présidente, madame la Ministre. Merci cher Annick de permettent de de prendre la parole sur ce sujet de la formation qui. Effectivement, est un sujet important, ça a été dit vous le tout tout le monde l'a rappelé ici on en a conscience. Je voudrais juste attirer votre attention et si vous pouvez transmettre le message au au ministre Pap Ndiaye. Su sur différents ce différents sujets le 1er c'est sur les personnels. Enseignants, vous l'avez dit, aujourd'hui, avec la massification de de l'inclusion chaque enseignant est confronté dans sa classe, ou le sera dans. Dans un cycle de temps très court à à la présence d'enfants en situation de handicap. Donc le, la formation des, des enseignants doit être. Doit passer à une autre échelle. Deuxièmement, c'est les personnels des collectivités. Parce qu'aujourd'hui on a la possibilité, voire même le. On n'a pas vraiment le choix d'embaucher les collectivités d'embaucher des personnels pour faire de cet accompagnement et aujourd'hui, eux, n'ont pas de formation ils ont pas de statut d'ailleurs un dans la fonction publique territoriale. À ESH donc ils sont adjoints technique ou adjoints d'animation et ils doivent avoir accès à la formation dispensée par l'Éducation nationale. Certes, certains. Certains rectorats le permettent. Mais n'informe pas ni les maires, ni les personnels. Donc on a besoin de cette information pour pouvoir inscrire ses personnels dans ces formations, et pouvoir Les et qui puissent être accueillis dans cette formation fait. Dispensés par l'éducation nationale. Et puis dernier point sur lequel je voudrais appeler votre attention, vous avez parlé de formation à la prise de poste ou formations continues c'est très bien. La formation est prise de poste, elle reste encore un peu inégal et et elles arrivent de manière très tardive dans la prise de poste parce qu'elle arrive dans la première année. Mais ça veut dire qu'on les envoie quand même pendant plusieurs mois devant les élèves sans aucune formation si on veut professionnaliser ce ce si on veut faire un métier de ces missions d'AESH en faire un métier, on a besoin d'une formation initiale, il faut qu'ils aient au moins une base de formation avant d'être en poste et ensuite bien sûr dans le cas de la formation continue, il faut approfondir cette formation et notamment de l'analyse de la pratique et qu'on puisse la différencier en fonction des de des cas des élèves qui qui suivent mais on a besoin d'une vraie formation initiale avant la prise de poste et puis je, j'insiste vraiment sur sur ce besoin de communiquer auprès des collectivités sur les offres de formation du ministère de l'Éducation nationale pour que les agents puissent y participer. Je vous remercie. Oui merci madame la présidente, bien entendu je vais je vais retirer comme le demande la rapporteure cet amendement et. Comme le disait à l'instant Cédric Vial, il ne peut y avoir de professionnalisation sans formation. Alors oui, madame la Ministre. Il y a des choses d'inscrite dans la loi, mais lorsqu'on voit que ces formations spécifiques, on comprend bien que dans les territoires formation spécifique c'est pas suffisamment précis et que cette application, hé bien géométrie variable dans nos territoires et ces auditions que je je reviens dessus parce que c'est vrai qu'au cours de ses auditions. On a vu des départements où ça se mettait en place mais d'autres où c'était absolument. Pas du tout. Mis en place avec des disparités à la fois sur la photo en formation initiale et continue, donc si tout ce qui était dans la loi été appliquée. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de travail s'est inscrit dans la loi mais on va rester mobilisés sur ce sujet parce que.

Nous avons fait des propositions. La mission. Le travail fait avec Marie-Pierre Monnier, Max Brisson. Donnait déjà des propositions pour des réponses donc emparez-vous de tout ce que tout le travail que nous avons pu faire avec la Commission d'éducation à la et et, culture et communication. Et puis on va pouvoir avancer parce que on n'a pas besoin encore de plusieurs mois pour établir les constats et les solutions je vous remercie.-- Même madame la présidente, que faites-vous de votre amendement suivant. Madame la présidente, comme vous avez pu le voir l'amendement. Suivant reprend la même thématique. Il est toujours question de formation. Je sais que de nombreux collègues aurait pu aussi déposé des amendements sur d'autres sujets. Il est question de formation et les questions de rémunération nous avons un un goût finalement de de frustration Madame la rapporteure sur ce texte mais nous savons que nous avançons d'un petit pas. Donc il va être demandé le retrait par ma collègue et rapporteur Marie-Pierre Monnier, j'accepte le retrait bien entendu je vous remercie. On va gagner du temps. C'était l'objectif de cette Merci. Si je vais donc ainsi mettre aux voix, l'article 1 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient été adoptée je mets aux voix l'article 2 qui est pour qui est contre qui s'abstient est adopté. Là tu supprimer, je vais mettre voilà l'ensemble de la proposition doit après avoir donné la parole pour les explications de vote.

Proposition de loi avec des auditions extrêmement intéressant et suivi par beaucoup de nos collègues, je voudrais remercier aussi les collègues parce que nous allons vers un vote conforme, donc on ne peut que s'en féliciter et c'est important aujourd'hui et j'ai une pensée pour Michèle Victory puisque c'est une PPL qui vient de l'Assemblée nationale et dont elle auteur. Je voudrais vous dire mais vous l'avez tous dit que oui cette proposition de loi est un 1er pas mais il faut le saluer. Et. De toute façon ce 1er pas nous engage à continuer à travailler le sujet sur le statut sur la rémunération sur l'organisation sur la formation cher Annick Billon, on en a beaucoup parlé, lorsque. On a eu des signes mais j'y reviendrai que le ministre voulait aller plus loin. Alors nous en sommes tout à fait conscient mais je voudrais aussi vous dire que cette proposition de loi est une reconnaissance et je crois que il faut le dire, de ces professionnels qui effectivement contribuent à l'école inclusive qui accompagne les enfants qui rassure les parents. Qui épaulent les enseignants. Je pense que c'est, c'est en tout cas extrêmement important dans la façon qu'on a eu aussi de travailler cette proposition de loi, alors on a senti que le ministre de l'Éducation nationale, vous voulez aller plus loin. Malheureusement et nous nous en félicitons. Malheureusement, il n'a pas donné de signe et singulièrement pendant la loi de finances où beaucoup de nos amendements sur les AESH. Eh bien ont été rejetés. Alors puisqu'il veut aller plus loin, il faut que avec le gouvernement Madame la Ministre il donne des gages. Très vite, que vous nous donniez des signes rapidement parce que vous avez vu que le Sénat est prêt à continuer et va continuer la réflexion va continuer le travail tout cas, c'est la volonté de beaucoup de collègues ici dans cet hémicycle. Alors cette PPL est une première brique allait à l'édifice. Mais je trouve que nous avons franchi une belle étape et à ce titre, je voulais vous vraiment tous vous remercier. Monsieur le président, la font. dans quelques instants, je l'espère à l'unanimité, évidemment il y a une petite frustration. Sur le fait que nous n'aimiez pas n'ayant pas pu l'enrichir les uns et les autres et que l'esprit de responsabilité, nous pousse à un vote conforme. c'est bien dans cet esprit que nous le faisons même si nous étions tentés, les uns et les autres d'aller au-delà, il faudrait pas du reste que ça prenne une habite que ça devienne une habitude. La peur de repasser dans dans un cycle de navette dans un contexte particulier qui est celui de l'annonce de l'Assemblée nationale, il ne faudrait pas que ça, ça freine les sénateurs dans dans leur initiative mais, parenthèse fermée. Moi je voudrais saluer bien sûr le travail de notre rapporteure Marie-Pierre Monnier. Notamment son constat. Qui a je crois réunis tous les membres. De la commission certainement mais aussi du Sénat. Constat qui est inquiétant. Inquiétant parce qu'on voit bien les efforts qui ont été faits et je ne, de ne les nie pas, notamment sur la montée en puissance. Du, du nombre d'AESH et l'organisation même si elle est imparfaite. Les efforts qui ont été fait côté État et côté Éducation nationale, mais malgré ça le le le résultat n'est pas encore satisfaisant, il n'est pas satisfaisant pour les familles et les enfants, il n'est pas non plus satisfaisant pour le personnel et en particulier les les les AESH donc je je crois que fort de ce constat. Il nous faut davantage encore travailler travailler avec l'État. Nous sommes assez bien sûr attentifs au à ce que vous êtes en train de faire, nous allons travailler de notre côté, à travers la mission de. Nous connaissons les forces et les faiblesses de l'éducation nationale nous connaissons cette capacité à monter en puissance à gérer 130.000 personnels. C'est certain nous connaissons aussi ses faiblesses et notamment. Les les disparités qu'on peut ressentir d'un territoire à l'autre, c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs parce que c'est un élément qui ressortait du constat de Marie-Pierre Le fait que d'un département à l'autre, la situation n'était pas la même et j'attire votre attention, madame la Ministre, sur ce point en particulier. Madame Jasmin. Merci madame la présidente, madame la ministre, j'ai une pensée à cet instant pour toutes les familles parce que là il s'agit aussi de réponse donnée à des familles. Donc je souhaite vraiment que vous puissiez aller plus loin. Bon j'adhère à tout ce qui a été dit avant. Mais depuis la loi de 2005, du 11 février 2005. C'est vrai que qui était déjà prévu l'inclusion en milieu scolaire et en milieu ordinaire des enfants justement une diversité d'handicap et beaucoup d'enfants ne peuvent jusqu'à maintenant pas aller à l'école parce qu'en fonction du type d'handicap et il y a pas forcément les réponses adaptées. Donc je souhaite vraiment à partir de maintenant que nous puissions collectivement travailler davantage à la fois pour répondre aux familles qui sont concernés et qui entendent aujourd'hui ce que nous faisons le travail l'avancée en quelque sorte mais aussi pour tous les AESH et là vraiment j'adhère également aux propos du chemin Billon parce que même si effectivement il y a des réponses dans la loi, mais on voit bien qu'il y a pas eu d'évaluation il y a pas eu non plus de réponses apportées jusqu'à maintenant à ces professionnels là où il faudrait vraiment qu'il y a un référentiel métier adapté pour que l'intégralité des handicaps et des personnes en situation de handicap des enfants en tout cas. Bénéficie des compétences de ces personnes et bénéficie également de tout ce que l'éducation nationale peut proposer à l'ensemble de ceux qui sont concernés. Je vous remercie. Madame Guillon. Oui merci madame la présidente. Donc le groupe Union centriste votera bien entendu le, la proposition de loi, c'est une première reconnaissance pour ces personnels à ESH et à ED. Qui vont peut être être plus facilement intégrer désormais dans les éduquer dans les équipes éducatives. Ils ont toute leur place dans ces équipes et il ne l'avait peut-être pas forcément donc ce ce 1er pas c'est c'est vrai véritablement à plus. J'ai souhaité insister sur la formation parce qu'il est question aussi de d'élèves en situation de handicap. Des élèves qui méritent une attention particulière, un accompagnement particulier et on ne s'improvise pas accompagnant lorsqu'on a des ondées handicaps et qui peuvent être très différents. Lorsqu'on doit accompagner des enfants pendant une semaine, qui ont des handicaps différents. Je voudrais aussi revenir sur la féminisation de de cette de cette profession de ces professions. On l'a dit, c'est essentiellement des métiers de femmes mais souvent lorsque les métiers se féminisent. C'était le cas lors d'une réunion de la délégation ce matin hé bien on voit que les conditions de travail, les conditions de rémunération se dégrade. Donc si nous pouvons-nous agir pour ce métier, qui sont extrêmement féminisés souvent exercée par des femmes. En situation difficile, parfois des familles monoparentales aussi avec des salaires qui ne permettent pas de de faire vivre une famille, nous devons le faire et c'est pas la rapporteure engagé dans la délégation aux droits des femmes qui me contredira. aussi sur ce que disait tout à l'heure notre collègue Françoise Gatel puisque au moment de la pause méridienne, un chef d'établissement m'a adressé un message. Sur la pause méridienne justement en me disant oui il y a cet avis du Conseil d'État du 20 novembre 2020. Alors les collectivités finalement à cette nouvelle décision, mais quid des établissements privés sous contrat. Qui n'ont pas parfois la même chance et donc qui qui qui vont peut-être favoriser des des des solutions alternatives qui sont pas satisfaisantes en terme d'égalité, donc c'est une question supplémentaire. Je vous remercie de m'avoir accordé ces quelques secondes supplémentaires. Madame la présidente. Merci. quelques mots tout madame la présidente, je vous je vous remercie. Juste pour dire que on on est très heureux de de l'issue probable désormais de ce texte et que je pense que c'est l'honneur du Sénat de montrer que sur des sujets comme celui-ci. Il peut y avoir un consensus qui traverse très largement tous les banques, quand on considère que c'est l'intérêt général avant l'intérêt partisan et cette proposition de loi qui vient du du groupe socialiste a été va être je l'imagine accepté dans des grandes proportions et et je m'en félicite. Deuxièmement, pour dire que c'est, avant tout, presque une carte postale au delà d'être ça sera une loi mais c'est presque une carte postale qu'on envoie ASH aux AESH pour leur dire qu'on que on on a conscience du problème et qu'on pense à eux par cette loi, permettre de faciliter ou d'améliorer la situation de quelques-uns. Mais le problème global il reste entier Madame la Ministre on vous l'a dit tout à l'heure, on compte beaucoup sur le, la réforme de à la fois du, du statut de la formation de l'accompagnement de manière générale du lien avec le médico-social avec la MDPH. Il y a un certain nombre de sujets qui reste vraiment à régler, on ne peut pas aujourd'hui gérer une organisation avec plus de 130.000 salariés. Sans avoir une organisation sans avoir un cadre. National ou un, ou un, un, un cadre de métier non madame, on pourra en reparler. Donc il faut vraiment remettre ce cadre là, c'est un sujet essentiel et on n'échappera pas non plus à la question que mon collègue Philippe mouiller a soulevé un peu tout à l'heure. Qui n'est pas qu'une question sémantique de savoir si le la ESH et dans un, un rôle d'accompagnement à la scolarité ou s'il est dans un rôle d'accompagnement au handicap c'est pas qu'une question de sémantique parce que derrière, juridiquement en termes de responsabilité et en terme de, de professionnalisation il y a aussi des enjeux auxquels je pense qu'il faut qu'on puisse en discuter et pour trouver les bonnes solutions. N'oublions pas que, au-delà il y a la question du statut des AESH mais il y a aussi derrière qui l'accompagnement nous voulons pour ses enfants dans dans l'école inclusive de de notre pays, je vous remercie. Merci madame la présidente, que la situation des AESH doit être considérablement améliorée, y compris après le vote de ce texte. Je suis particulièrement intéressé ce sont des débats que nous avons régulièrement en en commission de la culture. Notamment, mais je vois que beaucoup de nos collègues sont très sensibles au sujet et, notamment au sujet de la formation et je partage complètement ce qui a été dit sur la nécessité d'une formation initiale et continue et que la formation elle doit aussi intégrer les personnels enseignants pour que les AESH. Fasse mieux partie de la communauté éducative et soit reconnue à ce titre-là. Un dernier mot pour vous interpeller madame la Ministre, d'abord sur les rémunérations. Vous avez dit vous-même dans votre propos, vous avez rappelé vous-même que c'était là le 2ème. La La 2ème profession au sein de l'éducation. En terme d'effectifs et donc, ça n'est pas concevable que ses salariés soient encore même après. Les mesures de revalorisation prise en dessous du seuil de pauvreté. Et puis pour insister sur. Le fait que la possibilité ou offerte de laisser. Devienne une réalité parce que je le redis sur les à ED. Alors j'entends le décret, il a été pris cet été ce qui sûrement ne rendait pas les choses très aisé pour que les choses se réalise dès la rentrée, mais quand même à la lumière de ce qui s'est passé sur les à ED et le faible nombre qui ont bénéficié de l'aseptisation ont fait appel au gouvernement pour que vraiment des consignes soient données pour que ça se mette vraiment en oeuvre sur le terrain, je vous remercie.-- qui s'abstient. Elle est adoptée, je vais suspendre la séance pour quelques-uns. Elle sera reprise à 17h 40.

La séance est reprise. Pour la discussion de la proposition de loi visant à rétablir l'équité territoriale face aux déserts médicaux, et à garantir l'accès à la santé pour tous.

Madame la Ministre Madame la rapporteure chers en 1000 Houerou. Mes chers collègues je présente aujourd'hui devant vous. La proposition de loi que nous avons déposé avec notre collègue en 1000 Houerou et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain visant à rétablir l'équité territoriale. Face aux déserts médicaux, et à garantir l'accès à la santé pour tous. Déserts médicaux, ce terme est aujourd'hui sur toutes les lèvres, est au coeur des prix occupation de tous les Français. Nous connaissons les constats. Je n'y reviendrai que succinctement mais certaines réalités mérite néanmoins d'être rappelée ici. Aujourd'hui 11% des Français, 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant et parmi elles et essentiel. 657.000 personnes en affection longue longue 12 % de la population française vit en zone sous-dense et se dissuade situation, nous le savons va se détériorer dans les années à venir parce que les projections des effectifs établi par l'adresse font état d'une diminution des effectifs jusqu'en 2024 et un retour au niveaux actuels donc insatisfaisant seulement à l'horizon de l'année 2030. Ce contexte c'est d'autant plus préoccupant que la croissance démographique et le vieillissement de la population induisent une hausse toujours plus importante des besoins de santé.-- Je le dis en préambule ce texte n'a pas vocation à lui seul à résoudre l'ensemble des déchets, difficultés d'accès aux soins dans notre pays. La France connaît une pénurie profonde de médecins spécialistes comme généraliste les gouvernements successifs, soutenus par les syndicats et l'Ordre des médecins ont adopté dans une volonté de réduire les coûts de santé. Une politique de diminution de l'offre ainsi dans les années 70 nous formions 10.000 médecins par an, puis 3500 dans les années 90 nous informant aujourd'hui 1500. Nous avons voté il y a un plus de 2 ans numerus apertus dont l'efficacité, faute de moyens supplémentaires donnés à l'université pose aujourd'hui question à ce jour l'augmentation réelle du nombre d'étudiants admis en 2ème année de médecine est à peine de 10%. Nos politiques de santé, tout comme les études en médecine sont hospitalo-centrée et nous ont amener à négliger les politiques publiques notamment en une saveur de territoires ruraux. Aujourd'hui, les médecins sont issus des classes sociales supérieures et des métropoles, ce manque de mixité sociale et territoriale nuit à une répartition plus équilibrée sur le territoire. Nous avons fait beaucoup d'auditions rencontré de nombreux acteurs de terrain et face à cette problématique multifactoriel. Nous avons conscience qu'il n'existe pas de réponse simpliste facile ou même miracle mais que la réponse à cette problématique repose sur un ensemble de mesures coordonnées qui permettront d'améliorer de façon pérenne. L'accès aux soins.-- Notre conviction est aussi celle qu'une réponse aux déserts médicaux doit reposer sur un équilibre entre tous les acteurs, médecins, étudiants, collectivités territoriales et cetera qui chacun à leur niveau sont impliqués dans la santé des Français.-- La mise en place d'une année de profit d'une éducation Anne autonomie supervisée réalisé obligatoirement en zone sous-dense répond à la double ambition de meilleure reconnaissance de la spécialité de médecine générale et de lutte contre les déserts médicaux. Cette mesure permettrait de déployer rapidement 3500 à 4000 jeunes médecins dans les zones sous-denses, soit en moyenne 35 à 40 par département. les craintes exprimées par les étudiants et nous proposons ainsi de mettre en place une emmené de professionnalisation qui respecte les jeunes médecins les rémunère. À hauteur de ce qu'ils méritent et prennent en compte leur problématiques de vie cette année de professionnalisation ne sera donc pas un simple stage et sera et ses modalités de mise en oeuvre et en particulier une rémunération spécifique à la hauteur de leur parcours seront négociés, et j'insiste sur ce terme de négocier avec toutes les parties prenantes et en particulier les organisations syndicales des étudiants de 3ème cycle.-- Il est primordial pour que assurer l'effectivité de cette mesure qu'il y ait un réel intérêt pédagogique tendre sur la formation médicale elle-même que sur les modalités pratiques d'installation aussi cette emmener sera accompagné de l'encadrement pédagogique renforcé avec des médecins maître de stage universitaire. Cette proposition s'articule autour des départements échelle la plus appropriée selon le Haut Conseil pour l'amélioration de l'assurance maladie pour organiser la réponse en santé dans les territoires les étudiants choisiront donc leur futur lieu d'exercice sur une liste départementale fixé par une commission d'affectation et d'accompagnement à l'exercice de l'année de professionnalisation. Elle sera composée de représentants des universités de l'Ordre départemental des médecins de l'ARS départemental ainsi que d'élus locaux, les départements, comme c'est déjà le cas dans les Pyrénées Atlantiques avec présence 64 pour également gérer les conditions matérielles d'accueil des étudiants, ainsi que l'accompagnement dans l'installation définitive des jeunes médecins sur le territoire. L'exercice de la médecine a évolué et les jeunes médecins aspirent à un exercice en lien avec d'autres professionnels de santé. Néanmoins aujourd'hui encore un tiers des médecins généralistes exercent de manière isolée. Ce chiffre, bien loin des ambitions ma santé 2022 nous amènent donc à proposer de rendre l'exercice coordonné obligatoire dès 2026. Ainsi l'article 2 de notre proposition de loi défini une nouvelle organisation de soins centrés sur un partage des tâches entre médecin traitant et les autres professionnels de santé, au travers de protocole du établie par l'ensemble de l'équipe traitante cette équipe traitante sera coordonnée par un médecin généraliste, responsable du diagnostic et de et de la prescription et devra être la plus inclusive possible. Elle devra également être renforcées par des assistants médicaux et par des infirmiers de pratique avancée. L'exercice coordonné dans des équipes de soins primaires devraient être le plus souple possible et pour apprendre. Donc la forme le simple convention d'équipes de soins primaires ou alors une façon plus complexe. Les maisons de santé pluri-professionnelles ou les centres santé ainsi le partage des tâches, permettra de dégager du temps médical ce qui est essentiel et en priorité pour les patients sans médecin traitant ou en ALD à ce jour. L'exercice coordonné permis en outre une diversification de l'activité médicale exercice mixte avec un temps partiel en libéral, il a un temps partiel le salarié avec l'hôpital de proximité, la recherche ou la prévention institutionnel type PMI par exemple cela attire les jeunes. Pour répondre aux besoins de santé des territoires, nous proposons également dans notre article 3 de rétablir l'obligation de garde pour les médecins libéraux depuis 2002 et la décision du ministre Jean Jean-Max François Mattéi de supprimer l'obligation déontologique individuelles de garde. On observe une érosion de la permanence de soins 11 volontariat n'est pas suffisante pour répondre à la demande malgré les revalorisations financières régulières de l'astreinte. Seuls 38% des médecins, ils sont toujours les mêmes participé en 2021 à la PDS. Pendant les horaires de fermeture des cabinets, donc en particulier entre 20h et minuit ou le end, nos concitoyens n'ont comme seule ressource que d'aller à l'hôpital et cette situation participe bien sûr de l'engorgement des urgences hospitalières. Face au désarroi de la population qui se sentent délaissés. Il nous est paru. Indispensable de réinstaurer une obligation de garde par bassin de vie pour assurer la continuité de l'accès aux soins. Cette mission sera assurée en collaboration avec l'établissement de santé et en concertation bien sûr avec les professionnels.-- Depuis de nombreuses années les différents contrats d'aide à l'installation ont été multipliés. Pourtant malgré des sommes conséquentes. Le résultat n'est pas à la hauteur il nous sommes donc indispensable de mettre en place aujourd'hui une mesure forte de régulation à l'installation. Cette mesure vise à étendre aux médecins libéraux, un dispositif qui existent déjà pour d'autres professionnels de santé, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes l'adresse confirme que cette mesure apporte des résultats ailleurs dans le monde par exemple au Canada. Dans des zones donc qui seront définis par les ARS et en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un excédent en matière d'offre de soins. Un nouveau médecin libéral ne pourra s'installer en étant conventionnés à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cessera son activité. Loin de remettre en cause la liberté d'installation. Cette mesure a pour objectif de préparer l'avenir en orientant l'installation des médecins en fonction des besoins des territoires lorsque la démographie professionnelle permettra. Aujourd'hui, au regard de la pénurie et du nombre de médecins partant à la retraite dans les 5 ans. Cette mesure sera peu contraignante et l'entraîne pas comme certains le prédisent de vagues des content Enfin à l'article 5 nous visant à rééquilibrer les conditions de cotisations sociales des garanties de revenus et l'aide à l'installation qui doivent Venezi. De la même manière à la médecine salariée Calamity libéral. Les centres de santé sont souvent gérés et financés par des collectivités ou la Mutualité française et il convient de soutenir leur action en faveur de l'accès aux soins.-- Je conclurai en rappelant notre. Notre responsabilité collective. Comment pouvons-nous accepter le renoncement aux soins de nos concitoyens et la perte de chance que cela représente. Comment accepter aussi de renier notre promesse républicaine le droit fondamental à la ce détection de la santé et l'égal accès aux soins. L'accès aux soins étonnant le de santé publique et il est de notre devoir d'y apporter une solution.-- L'effondrement de notre système de soins, malgré l'implication de tous nos soignants mérite une grande loi santé mais celle-ci ne semble pas être à votre agenda Madame la Ministre ni même dans vos ambitions Nous vous proposons donc un texte volontariste pragmatique et rapidement opérationnel répondant à la préoccupation majeure des Français aussi si vous partagez cette ambition. Mes chers collègues, je vous demande de voter ce texte. parole.-- La parole est à madame Annie Le Houerou, rapporteur de la commission des affaires sociales.

Le groupe socialiste, écologiste et républicain a demandé l'examen dans son espace réservé de la proposition de loi que nous avons déposé avec notre collègue Emilia Ntoumi rôle visant à lutter contre la désertification médicale de nos territoires. Le constat connu et abondamment documenté je n'y reviendrai donc brièvement notre pays connaît de graves difficultés de démographie médicale qui sont appelés à perdurer par pour une décennie le temps nécessaire à la suppression du numerus clausus pour produire des effets et à la condition que le gouvernement donne réellement les moyens aux universités pour assurer. Ces formations. Les soins de 1er recours sont parfaitement affecté la France a perdu 5000 médecins généralistes, entre 2010 et 2021, quand elle gagnait 2 5 millions d'habitants sur la même période, l'âge moyen de la population française a augmenté de deux ans, tandis que la prévalence des maladies chroniques s'est accrue de plus de 2. L'inégale répartition des des professionnels de santé sur le territoire exacerbe encore davantage la difficulté. Les données récemment mis à jour par l'adresse montre que les 10% de la population les moins bien dotés ont accès en moyenne à une consultation médicale et demi par an et par habitant, contre une moyenne nationale de trois, quatre consultations par an. La qualification du territoire par les ARS retient que 72%. De la population vit en zone sous-dense. Il serait inutile de disserter ici sur les causes de cette situation et les raisons d'un tel défaut d'anticipation par les pouvoirs publics et les médecins eux-mêmes la responsabilité est partagée, il convient plutôt de trouver des solutions pour garantir aux soins sur des sous aux soins sur l'ensemble du territoire, dans l'attente d'un retour à meilleure fortune en en 2030. C'est à cette indispensable édifices collectifs que la proposition de loi entend contribuer. L'article 1er prévoit une année de professionnalisation à l'issue du DES DES diplôme d'études spécialisées de médecine générale afin de bien préparer les médecins à l'exercice de la médecine de ville, contrairement aux propositions déjà discuté il y a quelques semaines sur ces bancs, ce n'est pas une année de stage mais une année complémentaire d'exercice médical qui est ici proposé, elle sera assortie de conditions spécifiques visant à garantir son efficacité notamment par des conditions de rémunération négocier afin de garantir l'effectivité du dispositif cette année d'exercice. Son autonomie progressive sera réalisé à l'issue du 3ème cycle obligatoirement en en zone sous- dense. Il nous faut sur ce point, tenir un discours de franchise. Et assumer de demander aux diplômés une contribution de l'aide à l'effort collectif pour améliorer l'accès aux soins dans nos territoires. Pour favoriser la construction de projets personnels. Les jeunes médecins pourront librement choisir leur affectation sur des listes départementales établi en coordination entre les professionnels de santé, les autorités de santé et les élus, les élus doivent pleinement être reconnu dans. Ce rôle prendre leur part en créant des conditions d'accueil de qualité sur leur territoire et répondre aux besoins de logements d'accompagnement familial et personnel. C'est à cette condition que le dispositif favorisera l'installation en contrepartie nous souhaitons que cette année de professionnalisation enrichissent véritablement le parcours des étudiants et valorise justement l'effort demandé les jeunes médecins bénéficieront d'un statut spécial spécifique défini par décret après négociation avec les organisations syndicales, nous souhaitons qu'il se distingue nettement du statut d'internes et de Docteur junior et donne accès à une rémunération attractive.-- L'article 2 impose la constitution d'équipes de soins primaires avec d'autres professionnels pour l'exercice de médecine générale à compter de 2026. Il s'agit là de favoriser la coordination entre les professionnels de santé de 1er recours et l'élaboration de projets de santé répondant aux besoins des territoires.-- Ce dispositif n'a, n'a connu depuis 2016. Succès limité, seuls 220 ESP en cours ou en projet sont recensés par le ministère pourtant l'exercice coordonné constitue un outil indispensable non seulement pour structurer le parcours de soins mais aussi pour améliorer l'offre sur un territoire il accroît en effet l'attractivité de l'exercice en ville, surtout pour les jeunes médecins qui ne souhaitent plus s'installer de manière isolée, la tendance est. Il s'agit de l'amplifier. Pour gagner du temps dans sa mise en oeuvre.-- Pour mieux répondre aux attentes des professionnels. Le texte comporte les US conforte les ESP dans leur vocation de dispositifs souple complémentaire des maisons de santé. Centre de santé. T'es où communautés professionnelles territoriales de santé là CPTS en prévoyant que les équipes pourront consister en une simple convention conclue entre les professionnels. L'article 3 rétabli une obligation pour les médecins de participer à la permanence de soins.-- La permanence des soins ambulatoires la PDSA. Lorsque la. Continuité de ce service public l'exige. Le principe du volontariat individuel qui prévaut depuis la suppression de l'obligation de garde au début des années 2000 ne permet plus d'assurer une couverture satisfaisante de l'ensemble de nos territoires par la PDSA dans un contexte de démographie médicale déclinante et de désengagement. Il faut le dire de certains professionnels, il conduit également à concentrer l'effort sur les les médecins volontaires en 2021 d'après le ministère. Seuls 38% des médecins en moyenne participaient à la permanence, là encore, les inégalités se creusent entre les territoires. Le Conseil national de l'Ordre fait état chaque année de la progression des zones blanches et révèle que certains territoires ne sont plus couverts en soirée ou le weekend. Or la continuité de la PDVSA. Chaque fois que les besoins le justifie est indispensable pour améliorer la prise en charge des patients comme pour désengorger les services du d'urgence hospitaliers dont l'embolie. Encore été crainte l'été dernier et l'est encore à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est pourquoi le texte vise à renforcer en la matière la responsabilité collective des médecins en consacrant une obligation de continuité de la permanence sans rétablir pour autant un mécanisme disproportionnée et rigide de contraintes individuelles. Il ne conduit pas à imposer une obligation de garde à chaque médecin sans évaluation préalable des besoins, notamment en nuit profonde. Il appartiendra au contraire aux agences régionales de santé en lien avec l'Ordre des médecins et les représentants des professionnels de mesurer les besoins en soins non programmés pendant les horaires de fermeture des cabinets de définir en conséquence la permanence nécessaire et lorsque la continuité du service de justifie d'appliquer l'obligation dans chaque territoire l'article IV. Mais en place à compost un conventionnement sélectif dans les zones surdotées médicalement de telle sorte à ce qu'un médecin qui puissent être. Ne puissent être conventionnées que si ah praticiens déjà installés cesse son activité. Permettez-moi de répondre ici à quelques arguments régulièrement avancés pour refuser ce dispositif d'une pin nul ne prétend que ce mécanisme de conventionnement constituera le remède miracle pour orienter d'urgence, les médecins vers les territoires les plus sous-dotées. Le dispositif s'insère dans un ensemble de mesures incitatives et évite surtout que les déséquilibres territoriaux ne s'accroissent davantage d'autre part, il convient de récuser les reins. Les incriminations quant à une coercition excessive, bien au contraire. Les nombreux départs en retraite à venir le rendront rarement limitatif dans un premier temps. Il ne découragera nullement l'évocation médicale et les exercices conventionnés. En revanche, l'application de ce conventionnement conditionnel est de bonne politique publique elle anticipe le dynamisme attendu de la démographie médicale et prépare ainsi une installation équilibrée des promotions d'un terme plus importante. Enfin, l'article 5, propose que la distinction entre l'exercice libéral. D'une part et l'exercice salarié en centre de santé et d'autre part ne puisse suffire à fonder des différences dans l'octroi des aides conventionnelles visant à encourager l'installation des professionnels ou le maintien de leur activité dans des zones sous-dotées les conventions entre l'assurance maladie, les professionnels de santé prévoit toutes sortes de contrats incitatif aux paramètres variables. Il ressort de ce paysage confus que les aides ne sont pas systématiquement défavorables au Centre de santé cependant les contrats d'aide à l'installation des médecins sont clairement plus avantageux pour les médecins libéraux que pour un poste salarié en centre de santé. L'article 5 propose donc. De mettre fin à cette inégalité de traitement. Alors que les centres de santé concours aux côtés de la médecine libérale à l'accès aux soins de 1er recours dans les zones sous-dotées. vous l'aurez compris, mes chers collègues, à titre personnel, je suis favorable à cette. Proposition de loi, le texte prend acte de la pénurie de médecins et propose d'atténuer ses effets ils demandent pour cela des efforts proportionnés aux étudiants comme comme aux médecins et favorise l'indispensable coopération avec les autres professionnels de santé. C'est seulement par les efforts conjugués dans chaque territoire des pouvoirs publics, des professionnels de santé mais aussi dans une certaine mesure des patients que nous pourrons préserver l'accès aux soins partout sans concurrence néfaste entre les collectivités ou entre professionnels de santé. La commission des affaires sociales n'a toutefois pas adopté la proposition de loi. C'est donc le texte initialement déposé que nous nous apprêtons à examiner aujourd'hui. Je vous remercie. remercie. La parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la présidente, monsieur le vice-président de la commission, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs. À l'initiative du groupe socialiste votre assemblée examine cet après-midi une proposition de loi portant plusieurs mesures de lutte contre les déserts médicaux. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, comme ici au Sénat, les initiatives parlementaires se multiplient pour trouver des solutions face à cet enjeu clé pour nos concitoyens, celui de l'accès aux soins. Car le 1er des besoins le plus essentiel peut être et celui de l'accès pour tous et partout à la santé.-- Au delà d'être ministre. Je reste une professionnelle de santé et tous les jours jusqu'à ma nomination, j'ai pu constater comme vous les difficultés rencontrées par les Françaises et les Français à avoir accès à un médecin et se soigner correctement.-- Permettez-moi d'ailleurs d'être un peu taquine. Et de regretter que le gouvernement de François Hollande n'est pas jugé bon de supprimer le numerus clausus entre 2017, entre 2012 et 2017. Nous aurions gagné un temps précieux que nous n'avons plus aujourd'hui. Et pour mieux anticiper les évolutions de la démographie médicale. Et d'ailleurs peut-être que ceux qui aujourd'hui prônent l'obligation qui était aux manettes aussi entre 2002 12 et 2017 auraient pu le proposer. Car la situation, vous la connaissez, elle est préoccupante. 6 millions de patients sont sans médecin traitant dont plus de 650.000 en ALD. 87% du territoire français est aujourd'hui considérée comme une zone de sous-densité médicale des délais d'attente qui ne cesse de s'allonger une crise des vocations et une perte de sens pour le de nombreux personnels soignants. Devant cette situation qui n'est pas nouvelle mais qui s'est aggravée avec la crise sanitaire, le Plfss pour 2023 apporte de premières réponses dont une qui a recueilli l'assentiment de votre assemblée l'allongement à 4 ans de diplôme d'études spécialisées de médecine générale.-- Nous partageons donc pleinement votre volonté d'agir. Mais sur le fond, le gouvernement regrette les mesures de coercition, que vous portez dans votre proposition de loi l'obligation n'est pas la bonne solution. Nos voisins européens qui l'ont fait d'ailleurs en reviennent. Réguler le vide n'apportera rien et je ne crois pas que nous donnerons envie en obligeant.-- Ainsi l'article 1er de votre proposition prévoit de réaliser à l'issue du 3ème cycle des études de médecine, une année de professionnalisation obligatoirement en zone sous-dense. Nous partageons la volonté de mettre en place une 4ème année de professionnalisation mais nous divergeons sur la philosophie. Nous souhaitons plutôt inciter les étudiants en médecine à s'installer volontairement dans les territoires sous-dotés. C'est tout l'objet de la IV de la création de cette 4ème année de médecine générale dans le PLFSS dont le parlement vient d'achever l'examen. L'objectif est bien de donner confiance dans l'exercice ambulatoire, y compris en zones sous-dotées. La mission que François Braun et moi-même avons lancé sur la création d'une 4ème année de médecine générale a précisément pour objectif de travailler aux nouvelles modalités pédagogiques et aux modalités de répartition des terrains de stages et des praticiens maître de stage universitaire. Il s'agit bien de favoriser une affectation dans les territoires et zones sous-denses. Les dispositions prévues à l'article de vifs vise à rendre obligatoire l'exercice libéral de la médecine générale de premier recours, sous la forme d'équipes de soins primaires, lesquels pourront prendre la forme d'une convention entre professionnels de santé. Là encore, le gouvernement n'est pas favorable à l'obligation. Le risque d'une obligation à l'exercice coordonné au travers de ce dispositif et de ne pas réellement engagé les professionnels dans un projet collaboratif en rendant cette reconnaissance uniquement administrative.-- Par ailleurs, l'encouragement à l'exercice coordonné sous toutes ses formes. À l'initiative des personnels de santé eux-mêmes hé bien une priorité du gouvernement. Depuis mon entrée en fonction en juillet dernier. J'ai souhaité rencontrer lors de mes déplacements sur le terrain, les professionnels de santé qui ont fait le choix d'un exercice coordonné au travers d'une CPTS ou d'une ou J'ai ainsi rencontrer des structures qui fonctionnent bien.-- Mais aussi bien entendu d'autres qui fonctionne avec plus de difficultés. Toutes sont différentes mais celles qui fonctionne bien et cette heureusement la grande majorité ce sont celles où les professionnels sont pleinement à l'initiative.-- De même instauré, comme le prévoit l'article 3, une obligation à la permanence des soins obligatoires ne nous paraît pas adapté. Il est vrai que le taux de couverture en PDSA varie selon les territoires. La couverture des territoires par la PDA, ça n'est pas directement liée là aux zones sous-denses dans lesquelles les médecins participent le plus souvent la disparité de la couverture des territoires de PDSA pose la question de l'équité entre médecins ceux installés en zone moins dotée assurant nécessairement plus de garde de PDSA que les autres. Or la réintroduction de l'obligation individuelle de PDSA ne réglerait pas cette difficulté. Le principe de responsabilité collective, introduit par amendement gouvernemental dans le PLFSS 2023 nous semble préférable à un retour à l'obligation individuelle.-- L'article IV prévoit de soumettre le conventionnement d'un médecin dans les zones surdotées médicalement à la condition d'un médecin qu'un médecin déjà installés cesse son activité. Le gouvernement n'y est pas non plus favorable. Alors que la négociation conventionnelle est en cours. Nous n'entendons pas limiter de façon unilatérale la liberté de conventionnement des médecins en fonction de leur zone d'installation.-- Enfin, le gouvernement ne partage pas le bien-fondé de l'article 5. C'est bien. Je partage le constat que nous vous avez souligné dans votre rapport, madame la sénatrice sur la multiplicité des aides à l'installation, dont le nombre et les paramètres peuvent être source de confusion pour les jeunes professionnels, c'est bien dans cette perspective que le Plfss pour 2023 porte la création des guichets uniques d'accompagnement à l'installation des professionnels de santé ainsi qu'une simplification des aides données aux professionnels qui s'installeront.-- J'en viens au fond et la divergence que vous regrettez entre Centre de santé et médecine libérale. Ces aides conventionnelles fourni au centre de santé existe et relève des négociations conventionnelles entre les représentants des centres de santé et l'assurance maladie. Aujourd'hui les centres de santé peuvent être aidés à financer jusqu'à 3 médecins qui va longtemps plein sous condition que le centre de 100 santé, installé dans la zone sous-dotée reste ouvert pendant 5 ans et participe à la permanence des soins. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je me réjouis que nous ayons ce débat cet après-midi les défis et les attentes sur ce sujet sont immenses. Nous avons un devoir collectif.-- D'agir tous ensemble dans un esprit de responsabilité et d'engagement pour apporter des réponses concrètes et opérante aux besoins de nos concitoyens. Pour autant, et je conclurai par là l'instauration de mesures coercitives n'est pas la solution. C'est bien en partant des initiatives du terrain avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs et non pas contre eux que nous réussirons.-- Madame la sénatrice Pumerole. Je tiens à vous rassurer sur l'ambition

Dans la discussion générale. La parole est à madame Monique Lubin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.-- Madame la ministre. monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui porté par nos collègues Émilienne Miro. Houerou est le fruit du travail des sénateurs du groupe socialiste depuis plusieurs années maintenant. Nous avons déjà présentées, certaines de ces dispositions dans le cadre du débat parlementaire au cours de l'examen du texte et de propositions du gouvernement et d'autres groupes politiques qui nous ont semblé apporter des réponses insuffisantes à un problème de plus en plus aiguë. Nous sommes confrontés à une crise profonde et durable. Concernant l'accès aux médecins généralistes aussi bien que spécialiste. Nous l'avons rappelé lors de précédentes discussions dans les années 70, ce sont 10.000 médecins toutes spécialités qui étaient formés par an pour tomber à moins de 4000 en 2004 dont 2000 médecins généralistes, entre 8000 et 9000 dont 4000 généralistes, de 2011 à 2016 puis une nouvelle baisse des postes en dessous de 3400 de 2017 à 2021 pour les généralistes. Alors que la progression était continue pour les autres spécialités sur cette même période en 2022. Nous formons 9024 médecins dont 3634 généraliste. Une réduction de 67 et demi pour 100 en 50 ans dans ce laps de temps notre population est passé de 50 millions à plus de 65 millions d'habitants, soit une augmentation de 21% avec de surcroît la montée en puissance des problématiques du vieillissement de l'autonomie et de la dépendance. Ajouté au départ à la retraite des baby-boomers au chemin parfois long pour les médecins diplômés avant de pouvoir s'installer dans les territoires, ainsi qu'aux tensions liés aux multiples difficultés des secteurs du médico-social et de la santé. Sachant qu'il faut 10 ans pour former un médecin nous avons là les éléments d'une situation critique et nous en voyons les effets dans nos territoires. Qu'il s'agisse dans les Landes de Canning. Au Jean sous serre dans les Côtes d'Armor, de mon contours Bourbriac ou du Ménez ou en Haute-Garonne d'antichambre du Frontignan. Dorin ou de Bax. Et vous pourriez tous me citer des communes dans vos départements. Et ce malgré les efforts considérables accomplis par les élus locaux. L'adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale n'aura pas offert de réponse satisfaisante à ce problème. Il crée en effet une 4ème année d'étude pour les médecins généralistes sans rémunération prévue cette mesure reste très flou. Dès son annonce, elle a eu des effets délétères puisqu'un étudiant en médecine sur 3 à penser à arrêter ses études dans les dernières semaines selon une enquête de l'association nationale des étudiants en médecine de France parfois le remède est pire que le mal. Nous avons besoin de tout sauf d'une crise des vocations chez les futurs médecins. La France entre en tout état de cause, dans une période dans laquelle tout le territoire est ou sera en situation d'insuffisance chronique en matière de médecins. Le pays pâtit dément que des politiques de l'État que tout se paie aujourd'hui. Nos concitoyens qui sont confrontés à la situation angoissante de ne pas être assurés de trouver des rendez-vous médicaux dont ils ont besoin au péril de perte de chances de guérison et d'une grande réduction de leur qualité de vie. Les médecins eux-mêmes qui voient les listes de patients à suivre, s'allonger et ont plus que jamais besoin d'accompagnement pour assurer leur mission. Les élus locaux qui multiplie projets les innovations et les offres pour attirer les médecins sur leur territoire et les amener à s'y installer durablement dans une perspective de permanence des soins. Chacun de nous dans cet hémicycle, chacun de nos territoires et ou pour les plus chanceux sera concernée. La situation exige de nous. Des réponses qui apporte des améliorations sur le court, le moyen et le long terme et qui ne fassent pas plus de mal que de bien. C'est pourquoi au groupe socialiste, nous avons travaillé à partir de ces situations que nous constatons sur nos territoires relayé par ces vigies de la santé publique que sont aussi les élus. Nous avons auditionné et travaillé avec les associations d'élus, l'État, les représentants des médecins, et les syndicats de jeunes médecins. Nous avons oeuvré avec la conviction qu'il est aujourd'hui impératif de conjuguer une meilleure professionnalisation des médecins avec l'apport de temps médical dans nos territoires sous-dotés. C'est pourquoi nous avons investi à la fois le cadre pédagogique et l'apport de santé publique comme le soulignait dans cet hémicycle, notre collègue Bernard Jomier. L'une de nos propositions phares présentées dans cette loi est en effet l'année de professionnalisation dont nous avons déjà abondamment parlé ici. Elle a de nombreux avantages, au nombre desquels la reconnaissance et la rémunération à sa juste valeur de la contribution qui a demandé aux futurs et jeunes médecins. Elle prend également en compte leurs problématiques de vie en associant aux universités, les collectivités territoriales qui sont mieux à même de leur garantir des conditions matérielles adaptées en matière de logement, de transport et de vie quotidienne. Cette proposition de loi, si elle était adoptée, ne résoudrait pas à elle seule la crise des déserts médicaux mais elle apporterait des solutions opérationnelles qui se verrait tout de suite dans les territoires. Elle aurait le précieux Avantage de permettre de déployer très rapidement 4000 jeunes médecins généralistes, soit en moyenne 40 médecins par département. Notre texte bénéficier aussi grâce au travail d'une autre collègue Patrice Joly d'un article sur les conditions de l'exercice libéral et salariés. Notre proposition de loi a par ailleurs pour objectif de mettre en place une organisation du parcours de soin pour faciliter la prise en charge de chaque patient dans chaque territoire, cela sera rendu possible, grâce au gain de temps médical obtenu par une meilleure coordination entre les professionnels de proximité. Cette nouvelle organisation permettra de dégager du temps médical en priorité pour les patients sans médecin traitant et ou en ALD. Ce texte rétablira également l'obligation de garde pour les médecins libéraux pour permettre à la permanence des soins. Pour mémoire, la permanence des soins est un dispositif de prise en charge horaires de fermeture des cabinets médicaux depuis 2002 avec la suppression de cette obligation, on observe une dégradation du service rendu le volontariat n'est plus suffisant pour répondre à la demande. Il nous semble que cette voie que nous ouvrons est susceptible d'apporter des réponses d'ores et déjà concrètes efficace et pragmatique au problème des déserts médicaux qui nous taraude tous. Je vous remercie. La parole est maintenant madame Laurence Cohen pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, je veux remercier ici nos collègues Émilienne. Myrhol et Annie Le Houerou ainsi que l'ensemble du groupe socialiste pour le dépôt de cette proposition de loi qui vise à réduire qui vise à réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins qui ne cesse de se creuser dans notre pays, nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'en débat, tout dernièrement, d'ailleurs lors de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Contrairement au groupe les républicains et au gouvernement qui propose l'instauration d'une dixième année d'études de médecine en stage dans les déserts médicaux. Le texte propose l'instauration d'une année de professionnalisation obligatoire dans ces déserts médicaux. Il ne s'agit pas d'une simple incitation effectuer un stage dans un désert médical, mais d'une véritable année de professionnalisation avec un encadrement par un maître de stage universitaires et une rémunération à 3500 euros brut par mois. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit également que les modalités de mise en oeuvre devront être discuté avec les organisations syndicales des étudiants en médecine générale concertation qui était absent des propositions LR et du gouvernement face au manque de médecins généralistes. Le texte met en place une organisation coordonnée du parcours de soins de 1er recours. Nous ne pouvons rester dans une situation où 6 millions de nos concitoyennes et concitoyens se retrouve sans médecin traitant, y compris des malades en affection longue durée ces équipes de soins primaires sont une solution pour réaliser les actes de 1er recours par ailleurs la proposition de loi rétabli l'obligation de garde pour les médecins libéraux supprimée par le décret Mattéi de 2003 étant cette permanence de soins des établissements publics de santé aux médecins libéraux lorsque l'offre de soins du territoire de santé l'exige, notamment dans des disciplines comme l'ophtalmologie ou la radiologie c'est exactement ce que notre groupe porte depuis 2019 et notre proposition de loi qui a trait aux mesures d'urgence pour la santé et les hôpitaux de la même manière, nous partageons la nécessité de réguler l'installation des médecins dans les zones sur-denses comme cela existe pour d'autres professionnels de santé, notamment les pharmaciens, les infirmières, les orthophonistes, les chirurgiens dentistes, enfin la proposition de loi revient sur la disparité existantes entre les maisons et les centres de santé en matière de fiscalité, de conditions de cotisations sociales de garantie de revenus et d'aide à l'installation. Il est en effet inacceptable que l'aide financière accordée à l'installation des médecins libéraux et à l'installation des maisons de santé soit de 50.000 euros tandis qu'un centre de santé bénéficie d'une aide financière de seulement 30.000 euros. Je rappelle qu'à la différence des maisons pluridisciplinaires de santé, les centres de santé sont gérées par des organismes publics ou privés à but non but non lucratif et garantissent un accès aux soins de proximité sans dépassement d'honoraires et sans avance de frais surtout les professionnels exercent leur activité de manière salariés ce qui correspond à l'aspiration grandissante des jeunes médecins. En conclusion, cette proposition de loi qui reprend de Nemours. De nombreuses mesures comme je l'ai dit porté par notre groupe depuis de nombreuses années, va dans le bon sens à ces mesures d'urgence, il faudrait ajouter la suppression du numerus à part tu es prévoir d'augmenter des moyens des universités pour former davantage de médecins et par conséquent avoir une politique ambitieuse pour consolider consolider améliorer notre système de santé, de protection sociale mais c'est au gouvernement de prendre la main. En attendant, nous voterons bien sûr cette proposition de loi et j'en profite. Madame le Ministre puisqu'il me reste en un peu de temps de vous alerter après mon courrier. Adressé au ministre de la santé sur la situation des hôpitaux psychiatriques de Saint-Maurice ou ARS et direction ont prévu une opération immobilière de grande ampleur alors que psychiatrie et pédopsychiatrie sont en grande difficulté. Nous craignons avec mon collègue Pascal Savoldelli que ce projet purement spéculatif, porte un coup fatal à la qualité de la prise en charge des patients. Je vous appelle donc Madame la ministre à intervenir afin que la direction revoit sa copie. Je vous remercie. Merci.-- Bah, la parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste. Madame la présidente. Madame la rapporteure Madame la Ministre, mes chers collègues ma collègue Élisabeth Doineau étant souffrante je vais porter sa voix. L'accès aux soins et l'un des principaux sujets de préoccupation des Français aussi il est naturel que les parlementaires se saisissent de cette problématique et tente d'apporter des réponses par le biais de propositions de loi. Celle-ci se multiplient. Preuve que nous avons à coeur de répondre aux difficultés rencontrées en la matière par nos concitoyens sur tous les territoires. Le constat est largement partagée de nombreux rapports ont été publiés ces dernières années et les statistiques produites par des institutions comme l'adresse par exemple, permet d'appréhender en toute connaissance de cause, l'ampleur des difficultés. 2 raisons principales doivent cependant être redites le manque d'anticipation des pouvoirs politiques. Face au vieillissement de la population et le changement de la pratique médicale. Les jeunes médecins souhaitant légitimement aménager leur temps de travail avec leur vie familiale, d'un côté, un besoin de plus de temps médical pour plus de pathologies et de l'autre côté moins de temps médical par praticien. Cette proposition tente de répondre au problème de la désertification médicale. Je tente à mon tour d'expliquer pourquoi ces solutions ne sont pas les bonnes. Et pourquoi elles auraient même des conséquences préjudiciables sur notre système de santé et sur toute une profession. Je vais me permettre à titre personnel de passer sur l'article. Nous avons largement eu des débats similaires ces dernières semaines, en particulier à l'occasion du PLFSS. Concernant l'article 2 je n'y suis pas opposé sur le fond étant moi-même favorables à l'accélération du développement de la coordination entre les professionnels du travail pluridisciplinaire et en particulier à la pratique en équipe de soins primaires. Cependant, elle ne peut pas tout simplement se décréter elle nécessite la participation active des principaux concernés. C'est d'ailleurs ce que l'on observe dans la plupart des maisons de santé pluridisciplinaires et sur un plus large périmètre parfois quand il existe une CPTS cela demande du temps, de la volonté beaucoup d'investissement de la part de tous les professionnels de santé des paramédicaux jusqu'aux professionnels du médico-social. L'article 3 soulève le sujet essentiel de la permanence des soins ambulatoires elle recule fortement, ce qui accroît les tensions sur les services d'urgence hospitaliers néanmoins obliger les professionnels à assurer une permanence des soins dans un contexte de pénurie contribue à accélérer l'épuisement de ces professionnels dès lors que les rotations sont de plus en plus fréquentes, faute de relais. Attention donc à ne pas apporter une réponse plus néfaste que le problème initial. Enfin l'article IV pose le principe d'une arrivée de médecins conventionnés pour un départ dans les zones De l'aveu même de Madame la rapporteure. Cette mesure ne s'appliquera qu'à la marge.-- Quant à l'article 5. Certes, il est difficile de se retrouver dans le maquis des aides mais l'idée d'Annie lignée les aides pour les centres de santé à celle du MSP revient à encourager encore plus le salariat. Or, les chiffres ne montrent déjà cette tendance. Je n'y suis pas opposé en tant que telle mais l'exercice salariale diminue en moyenne d'un tiers le temps médical par rapport à l'exercice médical attention alors de ne pas l'accélérer davantage. Après ce réquisitoire, vous seriez tenté de me dire que la critique est aisée mais l'art est difficile. Quelle solution, alors je suis persuadé que nous avons déjà un arsenal d'outils mais que le plus difficile est de le mettre en oeuvre dégager du temps médical est ainsi possible en recrutant des assistants médicaux en répartissant le parcours de soins avec d'autres professionnels de santé, notamment des infirmières de pratique avancée, le partage des tâches est indispensable et logique il est parce que nous devons penser équipe traitante il est parce que la montée en compétence de certains professionnels de santé permet de répartir les prises en charge. Il est enfin parce que la coordination des soins, la complexité de certaines situations et la notion de parcours l'impose la télémédecine est aussi un outil qui a prouvé pendant la crise sanitaire. Combien il pouvait être utile lorsqu'il est bien encadrée. Je crois en la territoire autoréalisatrice des politiques de santé à chaque territoire, ses spécificités. Il conviendrait sans doute de déterminer une collectivité en charge de l'accès aux soins. L'échelon le plus pertinent et le département. Ce dernier avec l'ARS pourrait déployer des brigades de coordination et d'ingénierie pour accompagner les élus et les professionnels de santé sur le territoire de dernier point nous ne pouvons pas rester sourd aux demandes des médecins quant à la revalorisation du tarif des consultations qui est l'un des plus faibles d'Europe. Par ailleurs le PLFSS 2023, impulse un premier virage en faveur de la prévention mais un chantier énorme s'ouvre à nous d'une alimentation plus saine, à une activité sportive régulière en passant par moins de conduites addictives, plus de prévention c'est vivre en meilleure santé. C'est donc moins de besoins en temps médical. Améliorer l'offre en santé ne peut se résumer à ne traiter que la médecine de ville, il faut une refonte globale graduée entre la ville et l'hôpital. Le gouvernement a lancé les travaux du Conseil national de la refondation sur la problématique santé attendons ses conclusions et les 2 actions qui en découleront. Pour conclure, je crois qu'il convient d'assumer un discours de vérité. Nous savons que la prochaine décennie sera encore difficile. La régulation, c'est une coercition qui ne dit pas son nom et ça ne elle ne répondra pas à la pénurie. À l'inverse, la coopération peut nous aider à passer ce cap difficile. Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe Union centriste ne votera pas cette proposition de loi. Je vous remercie.--

Monsieur il a décidément aujourd'hui Madame la rapporteure, chers collègues, cette proposition de loi pose un constat partagé sur tous les bancs de cet hémicycle, nous observons en effet depuis plusieurs années un recul de l'accès aux soins et un déclin de la permanence des soins. Ces sujets sont une préoccupation voire une inquiétude grandissante pour les élus patients et professionnels de santé, les chiffres le confirment, en 20 ans, nous avons perdu 18% de généralistes 9% de spécialistes hein bon nombre d'entre eux vont partir à la retraite alors que les besoins liés au vieillissement de la population et à la prévalence des maladies chroniques augmentent et que les jeunes médecins. Cela a été dit, comme le reste de la population d'ailleurs son. Et c'est légitime de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Nous avons donc un problème, un problème de pénurie. Bien plus qu'un problème de répartition. Cette pénurie a été instauré dès le début des années 80 à des fins. De régulation de dépenses de santé, il fallait boucler à l'époque, le trou de la Sécu, comme en témoigne le slogan des années 90, la Sécu c'est bien, en abuser ça craint. Tous les gouvernements de droite et de gauche ont poursuivi cette mesure mortifère pendant plus de 2 décennies. Voilà la principale raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et que patients et professionnels subissent au quotidien. Alors l'augmentation du numerus clausus puis sa transformation numerus apertus décidé tardivement. Vous l'avez dit Madame la Ministre ne porteront leurs fruits que dans une bonne dizaine d'années à ce sujet pouvaient pourrons-nous avoir des chiffres précis sur le nombre d'étudiants entrés en médecine et notamment en médecine générale sur ces dernières années, combien de médecins supplémentaires. Pouvons-nous espérer pour 2030 et seront-ils en nombre suffisant pour faire face aux enjeux qui nous attendent demain. Face à la pénurie. La PPL que nous examinons propose encore de renforcer les contraintes et les obligations à l'article premier stage obligatoire dans les déserts médicaux à l'article 2, obligation de création des équipes d'équipes de soins primaires, à l'article 3, obligation de garde à l'article IV régulation à l'installation. Or nous devons tous prendre conscience qu'aujourd'hui, la médecine générale n'est plus attractive et je crois que ce ne se là n'est pas assez dit. Pour preuve, elle est l'avant-. Dernière spécialité au classement du classement aux épreuves nationales classantes, fameuse au CN et les raisons sont multiples contraintes administratives, charge de travail grandissante perspectives de carrière limité en effet fini l'accès au métier d'urgentiste de gériatres, fini les diplômes universitaires dans géologie ou de médecine esthétique qui permettait de diversifier la la profession suppression du stage libre des ça se passe une quatrième année que l'on a failli encore limité à la pratique ambulatoire les tentatives répétées et nombreuses de renforcer les obligations pour régler plusieurs décennies de politiques publiques de santé défaillante, ne réconcilieront pas les jeunes avec l'exercice de la médecine générale, les professionnels font face à des conditions de travail suffisamment dégradée. Je ne crois pas qu'il faille les aggraver en faisant peser davantage de contraintes sur ceux qui tiennent tant bien que mal, notre système de santé à bout de bras. C'est avec eux et pas contre que les solutions seront trouvées notamment dans le cadre de négociations conventionnelles qui sont en cours avec l'assurance maladie. dans ces négociations conventionnelles. Il faut miser sur la responsabilité collective, notamment dans la PDSA. Vous l'aurez compris, nous ne croyons pas que les mesures proposées par cette PPL puisse résoudre nos problèmes en période de crise et de pénurie en attendant que le numerus apertus produit ses effets, nous devons au contraire serrer les rangs instaurer la confiance. Laisser le terrain s'organiser comme il a su le faire pendant la crise Covid décharger les professionnels des tâches administratives valorisé respecter leur travail lever les freins et accélérer le déploiement d'outils déjà existants. Je veux parler MSP ou toute forme d'exercice coordonné l'assouplissement des règles de cumul emploi-retraite les assistants médicaux, les infirmières de pratique avancée ou encore le déploiement de la télémédecine, voir le partage de tâches pour in fine donner envie aux jeunes de s'engager dans cette voie. Je crois que ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons améliorer l'accès aux soins partout et pour tous, pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette PPL.

Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues. Madame la rapporteure j'interviens en lieu et place de notre collègue Jean-Claude en glace, sénateur de l'Aveyron, je le précise bien, vous comprenez tout à l'heure pourquoi. La désertification médicale n'est pas un problème récent. Environ 30% de la population vit dans un désert médical chiffre qu'il faudrait encore précisé selon les spécialités. Les constats sont connus, ils ont été rappelés. Je ne reviendrai pas sur le sujet. Dans le contexte actuel où la question de la juste rémunération de l'acte se pose de manière accrue. Étendu que la désertification médicale ne porte pas seulement sur la médecine générale qui serait donnera nécessaire de penser la question de l'inégalité d'accès aux spécialistes, et à d'autres patricien cette proposition de loi Robien sous des débats que nous avons déjà eu au Sénat. Mais d'abord pas de nouveau sujet. L'instauration d'une année de professionnalisation obligatoire dans les déserts médicaux pour les médecins généralistes en fin de formation renvoie à des débats très actuel, de même que l'objectif d'une meilleure reconnaissance de la spécialité de médecine générale. Par ailleurs, l'idée d'une départementalisation des affectations mériterait d'être étudié dans le futur pour lutter contre les déserts médicaux. Même si le cadre géographique des centres universitaires et évidemment la région autour des Cependant, cette proposition de loi comporte des éléments à satisfaisant. J'en tiens avez IV. D'abord, contrairement à la proposition de loi adoptée le 18 octobre dernier visant à la consolidation et la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale, celle que nous examinons aujourd'hui ne prévoit pas d'en faire une spécialité à part entière.-- Ensuite c'est l'obligation de garde pour les médecins libéraux est un facteur pour désengorger les urgences médicales. Il ne me semble pas nécessaire de devancer voire de sur planter les discussions en cours entre la profession et les autorités de tutelle. Enfin, le dispositif de régulation à l'installation et celui du rééquilibrage des cotisations sociales des garanties de revenus et de l'aide à l'installation entre médecins libéraux et salariés ont déjà été discutés et rejetés lors de l'examen du PLFSS, pour des raisons pertinentes. Plus largement cette propositions de loi comme d'autres ont à s'inspirer plus ou moins des solutions trouvées dans certains territoires. Il y a des enseignements à tirer des expériences locales. perspective perspectives j'évoquerai les facteurs de la réussite de la politique d'attractivité expérimenté on Aveyron depuis 2010 pour inciter les médecins de médecine générale à s'installer. Dans le contexte d'un département rural du Massif central, caractérisée par un vieillissement de la population et un éloignement des urgences et des hôpitaux. La permanence des soins de proximité du maillage territorial en médecine générale a été un préalable essentiel pour penser le problème de manière globale à l'échelle d'un territoire. En ce sens avec le concours du Conseil de l'Ordre des médecins de l'université de Rangueil, ainsi que de l'ARS départemental d'une part, nous avons développé l'accueil des stagiaires pour faciliter l'implantation sur le territoire. D'autre part, nous avons été précurseurs soit l'approche d'organisation collective en maison de santé pluridisciplinaire et en réseau de santé. L'efficacité et le succès de cette organisation auprès des professionnels. Oh, conduit à la labellisation en CPTS la première CPTS en Occitanie et peut être parmi les premières de France. Ainsi, il est nécessaire de répondre aux envies aux besoins des jeunes praticiens qui ne veulent plus être isolé. Le partage des tâches et la coordination avec les autres praticiens sont au coeur des nouvelles pratiques afin de favoriser l'installation sur le territoire.-- Le développement des stages en Aveyron et le statut du médecin maître de stage ont favorisé la transmission et la sédation de jeunes médecins. La formation médecin sapeurs-pompiers à destination des internes a aussi renforcer l'intégration. Le succès de la lutte qu'aurait DiDomenico repose enfin sur un accompagnement concret à l'installation.-- 14 ans après les premières mesures en Aveyron. 9% de l'effectif des internes. Il reste à l'issue de leur stage, contre 1% en moyenne pour les territoires ruraux. Depuis 2011 il y a eu 105 l'assaut de médecins généralistes pour 107 départs, soit un renouvellement de l'effectif. Certes l'Aveyron est beau mais cela ne suffit pas à expliquer cette réussite. Celle-ci reposent plus certainement sur la mise en place d'écosystèmes qui font émerger des conditions favorables à l'intégration de nouveaux praticiens. cette proposition de loi arrive trop tôt parce que la concertation entre les professionnels de santé et les pouvoirs publics dont nous avons parlé, est toujours en cours et elle arrive trop tard parce qu'elle reprend les débats que nous avons déjà eu. Comme mes collègues du groupe LR, je ne voterai con contre cette proposition de loi.-- Merci ma parole est maintenant à Monsieur Daniel Chassain pour le groupe les indépendants. Madame la présidente, madame la ministre madame le rapporteur. Monsieur le président, mes chers collègues. Le sénat examine ce soir un nouveau texte pour lutter contre les déserts médicaux. Ce texte poursuit le même objectif que la proposition de loi de loi du président Bruno Retailleau et que le projet de loi de finances de financement de la Sécurité sociale. Cette proposition de loi arrive. On peut dire à contretemps. Et pourtant le problème qu'elle soulève reste entier. Une autre initiative transpartisane vient d'être présenté à l'Assemblée nationale le Parlement reste mobilisés notre groupe considère qu'il est important que le Sénat puisse débattre de ces enjeux. Qui affecte tout particulièrement nos territoires ruraux. Merci à notre collègue des moules Émilienne Pumerole. Le déficit chronique des Médecins de France. En France, c'est le résultat de plusieurs décennies d'inaction. Le remplacement du numerus clausus par le numerus apporte va dans le bon sens, mais bien sûr pas assez rapidement. L'article 1er. De ce texte vise à ajouter une année de professionnalisation dans le cursus de formation des étudiants médecins généralistes cette année devrait devrait être réalisé dans un désert médical en pratique ambulatoire auprès de maîtres de stage universitaires. Cette mesure va d'un bon sens je crains pour ma part quelle condition liées à l'encadrement du stagiaire par un maître de stage universitaires universitaires soit parfois contreproductif. En effet il être difficile de trouver partout des maîtres de stage, surtout dans certains départements, loin des CHU. C'est pourquoi je proposerai 2 amendements afin d'assouplir les conditions en prévoyant. Qu'une année où six mois au moins. Puisse être réalisée auprès d'un médecin traitant référent l'exposé des motifs de la proposition de loi indique que les étudiants pourront toucher 3500 euros nets par mois, j'avais proposé pour ma part une rémunération équivalente à 10 consultations par jour, soit 5000 euros par mois ce revient cela revient peu ou prou la même chose car il y a des frais de voiture je tiens à dire que l'organisation de ce système en lien avec le conseil départemental et pour moi pertinent le département et la collectivité de proximité, la plus adaptée. Les conseillers sont proches des maires et connaissent la réalité du territoire. L'article de ces prôner la coordination entre les professionnels bien sûr c'est bon. Et la la MSP le favorise. L'article 3 de de la proposition de loi rétabli l'obligation de garde pour les médecins libéraux. Notre groupe, c'est que cette mesure est contraignante et peut nuire à l'attractivité du statut cependant elle nous paraît nécessaire pour garantir l'accès aux soins partout en France, le recours aux CPTS, nous sommes bien sûr pertinents. L'article 4, quant à lui. lui. Instaure un conventionnement sélectif c'est-à-dire prévoir que médecin libéral ne peut être conventionnés en zone dense, sauf si l'un de ses confrères déjà installés cède sa place. Nous y sommes favorables. Elle répond à un besoin exprimé par de nombreux élus des territoires ruraux. En revanche, l'article 5 de cette proposition de loi pose un problème. Cet article prévoit une égalité de traitement en matière d'aide publique entre médecins libéraux et médecins salariés or les conditions d'exercice des médecins salariés et libéraux ne sont pas les mêmes. il faut être clair, les médecins salariés ne peuvent pas garantir une offre de soins complète sur l'ensemble des territoires. Il existe trop de contraintes d'organisation liées au droit du travail. Le salariat répond peut-être aux aspirations de certains jeunes médecins c'est peut-être possible dans à l'hôpital où il y a mais les médecins libéraux prodigue. Plus de présence de soins que les médecins salariés ils sont donc les plus à même pour lutter contre les déserts médicaux et je rappelle qu'ils gèrent ensemble avec les paramédicaux, les maisons de santé dans un 4 associatif, c'est pourquoi je vous proposerai un amendement de suppression de l'article 5. Cette proposition de loi a le mérite de remettre dans le débat. Un sujet d'extrême importance pour la cohésion territoriale et sociale de notre pays, notre groupe se déterminera en fonction des ajustements proposés. Je vous remercie.-- Merci la parole est à Madame. Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste solidarité et territoires.--

Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, chers collègues. C'est la deuxième. Vois ces derniers mois, que nous débattons du sujet prégnant des zones sous-denses, preuve de l'urgence de la situation et du manque de réponses à la hauteur du gouvernement. Le constat est connu et s'aggrave un médecin sur 2 ne prend plus de nouveaux patients alors que 660.000 patients en affection de longue durée n'ont pas de médecin traitant quasi générale ne doit pas masquer des disparités entre territoires qui s'approfondissent car 30% de la population vit dans une zone d'intervention prioritaire, zone fortement Les zones rurales sont particulièrement touchés et subissent le non remplacement des médecins conjuguée à la fermeture des hôpitaux de proximité, des services d'urgence. Ou des maternités. En conséquence, 60% des personnes en territoires ruraux ont des difficultés d'accès à un médecin généraliste selon l'adresse et 6 millions de personnes se retrouvent sans médecin traitant, particulièrement les jeunes mais aussi les pauvres et les plus isolés. Devant ces inégalités territoriales qui se creuse. Nous avons le devoir d'agir et vite car la fin du numerus clausus pour autant qu'il serait suffisant ne portera pas ses fruits avant une décennie ce qui oblige à gérer le moyen terme, via par exemple comme le propose cette PPL des mesures plus contraignantes de planification de l'offre. Car jusqu'à présent les mesures d'incitation financière se sont soldées par des échecs et comme pointée par la Cour des comptes, elles ont plutôt provoqué des effets d'aubaine pour des médecins exerçant déjà en zone sous-dense. Face à cela le gouvernement ne propose que des demi-mesures pour ne parler que de la mesure du PLFSS sur la dixième année certaines études concluent en effet qu'un stage long en zones sous-dotées peut encourager certains médecins à s'y installer. Mais qui peut croire qu'il s'agirait là d'une solution suffisante. Pour notre part, d'ailleurs nous pensons que le 1er site devrait être raccourcie et qu'il est dommage qu'une dixième année soit ajouté sans refonte de l'ensemble des cycles en tout état de cause, la volonté qu'elle se fasse prioritairement en zone sous-dense ne peut s'entendent que si parallèlement.-- Des mesures de régulation s'applique à tous les professionnels et pas seulement aux jeunes médecins entre. Nous sommes donc assez favorables aux autres mesures de régulation équilibrant l'effort. Ainsi de conditionner le conventionnement des médecins en zones surdotées ont remplacement à l'identique sur le territoire de vie santé concernés pour ne pas accroître encore les inégalités. Et ce, à l'instar à de multiples autres pour de multiples autres professionnels de santé. Tout comme la mesure l'établissement rétablissant par la responsabilité collective. L'obligation de participer à la permanence des soins ambulatoires car aujourd'hui ce ne sont plus que 38% des médecins qui participent. On l'a dit, mais contre 67% il y a 7 ans avec de fortes disparités territoriales et ce chiffre ne cesse de baisser. Voilà le résultat du laisser-faire et de l'appel au seul volontariat. Mais ces mesures doivent s'inscrire dans des réformes structurelles qui engage aussi le long terme. En l'occurrence pour réduire les déserts médicaux. La solution passe aussi par la décentralisation des premières années de médecine comme le recommande l'OMS comme amorcé timidement en France et de la et de la diversification des étudiants. Car selon la méta-analyse de l'adresse. L'origine géographique et social des étudiants ressortent dans tous les pays, comme des déterminants majeurs du choix d'installation. Ah si, être originaire d'une zone rurale accroît l'intérêt d'exercer en zone rurale, souvent très dans Parallèlement donc à ces réformes structurelles que nous appelons de nos voeux ce texte propose dès maintenant des solutions de régulation et c'est pourquoi le groupe écologiste votera pour. Je vous remercie. La parole est au président du groupe RDPI François Patriat. Madame la présidente, madame la ministre madame le rapporteur Monsieur le dicton de la commission. Mes chers collègues.-- Chercher désespérément un rendez-vous médical de voir se rendre aux urgences, faute de médecins disponibles. Nous avons tous pour beaucoup d'entre nous vécu ces moments de désolation. Face à un système de santé parfait. Quand l'accès aux soins devient un parcours du combattant, il faut agir. Comment parvenir demain à ce que chacun puisse avoir accès à un médecin proche de chez lui et rapidement. Pour y répondre, les propositions sont multiples mais face à cet éventail de choix il faut trouver un juste équilibre entre coercition et laisser faire entre incitation et obligation entre belles idées réalité, les choses sont plus complexes. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui soumis propose une version très coercitive 4 articles.-- Donne des obligations impôts des obligations obliger les médecins généralistes à réaliser leur année de professionnalisation dans des zones sous-dotées obligé une organisation de professionnels de santé en équipe de soins primaires à partir de 2026 obliger les médecins libéraux réaliser des gardes obligé d'une certaine manière les médecins libéraux à s'installer dans des zones précises et l'obligation comporte plus de risque. Celui de voir nos futures générations de médecins privilégier l'existe le mais l'exercice salarié plutôt que l'exercice libéral, celui d'une fuite des professionnels de santé, vers l'étranger, où les propositions ne manquent pas. Le risque enfin que les médecins libéraux qui se plie à ses obligations se voient submergés sous les demandes avant les effets de la suppression du numerus clausus et quelques médecins installés en zones sous-dotées qui se partageront le poids des gardes risquerait alors le surmenage. Mais ce n'est pas acceptable que nos citoyens, nos concitoyens ne parviennent pas dans certaines zones à trouver un médecin disponible en soirée et se aux urgences parfois loin de chez eux pour des raisons qui n'en sont pas. Il n'est pas acceptable que certains de nos territoires se voient privés de médecins et que nos concitoyens se retrouve esseulé face à des pathologies complexes. 11% des Français de plus 17 ans n'ont pas de médecin traitant. Un million, 6 Français renoncent chaque année aux soins médicaux. qu'il faut répondre à cette situation et tout en sachant, comme l'a montré le titre du CHU de Clermont-Ferrand. De quelques années, 45% des médecins généralistes français exerçant en libéral était en situation de burn-out alors aller contre la volonté des médecins ne me semble pas le plus productif. Face à cette situation. Des mesures fortes ont déjà été prises, telle que la suppression du numerus clausus. On a dit l'exonération des cotisations de retraite pour les médecins libéraux en cumul emploi-retraite pour 2023. La notion d'une responsabilité collective de participation à la permanence des soins. Cette dernière étendu aux chirurgiens dentistes, infirmiers diplômés d'État et puis aux sages-femmes. L'expérimentation pour permettre des consultations de médecins généralistes et spécialistes dans des zones sous-dotées. Je crois qu'il faut le laisser le temps à ces nouvelles mesures de prendre effet si la responsabilité collective ne suffisait pas. Alors oui le rétablissement des gardes obligatoires s'imposerait mais donnant le temps à la concertation. On pourrait par exemple demander à ce que les gares soient faites de 5h à minuit. Après c'est l'urgence absolue 5h à minuit mieux rémunérés avec des hôpitaux qui enverrait pour les week-ends où sont en zones sous-dotées des médecins ou des internes de garde qui pourrait assurer ces gardes localement. Plusieurs autres pistes de réflexion ont été proposés par nos collègues Patricia Schillinger et Philippe mouiller dans le rapport. Renforcer les Liens entre les collectivités et la faculté de médecine utiliser davantage la télémédecine, ou encore renforcer le déploiement de contact de contrats locaux de santé sans être une solution unique. Ces mesures pourraient être des outils pour répondre à l'enjeu d'égal accès aux soins. La concertation ne semble être la voie privilégiée. C'est tout l'objet de CNR territoriaux sont en cours, j'étais moi-même présent à la semaine dernière à celui de Dijon et en échangeant avec des professionnels de santé, nous pouvons voir que nous souhaitons tous une amélioration de l'accès aux soins, une meilleure répartition entre médecine de ville et l'hôpital, une plus grande coordination entre les professionnels, alors que le but est partagée, il semble préférable de chercher ensemble des solutions grâce à une concertation et sans décourager les médecins libéraux. Alors, mes chers collègues compte de 30 tenu du fait que le texte est trop contraignant et que pour notre part nous reprendre. Nous sommes en mesure de retenir plutôt la possibilité de restaurer un système de garde obligatoire, nous nous abstiendrons sur le texte, je vous remercie. Merci. Madame Corinne Imbert et la dernière oratrice de cette discussion générale pour le groupe et l'intérêt

Madame la présidente, madame la Ministre, Monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous discutons, nous discutons donc aujourd'hui de la proposition de loi visant à rétablir le. Les quitter territoriale face aux déserts médicaux, et garantir l'accès à la santé pour tous. Ce sujet fait régulièrement l'objet de propositions de loi de rapports de diverses questions à l'initiative des sénatrices et sénateurs et a occupé une partie de nos débats lors de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En effet l'accès aux soins demeure un sujet de préoccupation essentielle chez nos concitoyens et chez les élus locaux. La réalité, nous la connaissons tous au sein de cet hémicycle, nous partageons les constats. Mais le manque de médecins généralistes ne touche plus seulement de campagne mais également constatée dans de grands centres urbains je dirais urbains et ruraux tous ceux concernés. Les raisons qui ont conduit à cette situation sont multiples. Et le problème plus complexe qu'il n'y paraît. Les élus locaux se sentent désarmés face à cette situation et de compatriotes demeure dans le désarroi le plus total lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés en matière d'accès aux soins. Mais nous n'en serions peut-être pas discuter de la création d'une année de professionnalisation pour les médecins généralistes en fin de formation. Si le gouvernement avait pris le décret d'application de la disposition votée dans la loi Santé de 2019 à savoir au moins six mois en troisième année d'internat de médecine générale en autonomie supervisée auprès d'un médecin généraliste en zone sous-dense. Un décret d'application jamais pris, malgré les promesses des ministres dont acte. Mais notre système de santé suffisamment mise à mal, y compris sur le plan éthique et je vous renvoie, mes chers collègues, à la vie 140 du comité consultatif national d'éthique qui qui vient juste d'être publié tout récemment pour que ce défaut d'application d'une loi soit tu acceptable, je souhaite que le gouvernement Madame la Ministre prennent la mesure de cette insuffisance, en particulier sur les sujets et les textes relatifs à la santé. Mais revenons au texte. L'article 1er de cette proposition de loi instaure donc une année de professionnalisation à la suite du 3ème cycle de médecine générale. Loin d'être opposé à cette mesure. La majorité sénatoriale. Adopté en octobre dernier, la proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation en médecine générale, déposée par le président Bruno Retailleau. Cette proposition de loi prévoit que le 3ème cycle de médecine générale sera d'au moins 4 années comme l'ensemble des autres spécialités. Plus solide sur le plan législatif, nous privilégierons sa rédaction. Même si l'objectif de chacune de ces propositions de loi peut se rejoindre. L'article 3, vise à rétablir l'obligation de garde pour les médecins libéraux. L'article 4 vise à étendre aux médecins libéraux, un dispositif de régulation à l'installation. Notre famille politique est historiquement attachées au caractère libéral de la médecine de ville, il apparaît illusoire d'évoquer en 2022. La notion de zones surdotées cela a pu être le cas par le passé mais cette notion apparaît aujourd'hui comme dépassé. Alors que le temps médical est compté. Nous ne sommes pas certains des effets supposés bénéfiques de cette mesure, ou tout du moins nous pensons au contraire que ces effets collatéraux seront largement sous-estimé notamment en termes d'attractivité pour la médecine générale.-- Enfin et surtout, et cela a déjà été dit, à l'heure où des négociations conventionnelles se sont ouvertes entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins pour une durée de 6 mois, il apparaît primordial de garantir la sérénité de ses dialogues au cours duquel je n'en doute pas les points abordés par les articles 3 et 4 seront discutées. Le vote unilatéral au Sénat d'une mesure coercitive à l'installation serait un mauvais signal envoyé nous préférons attendent les conclusions des négociations conventionnelles. L'article 5 concernent Centre de santé. Nous estimons que les médecins libéraux et des médecins salariés n'ont pas les mêmes contraintes à ce titre ils ne doivent pas être aidés de la même façon la réalité ce que les centres de santé ne sont pas la solution idéale. Certains centres de santé n'arrive même pas à recruter la totalité du nombre de 1005, il s'était fixé et une aide un médecin salarié ne doit pas être une subvention déguisée. Un centre de santé, il faut bien si nous reconnaissons tous ensemble qu'au début de leur fonctionnement, ils sont souvent déficitaires. En face, qui a rappelé que la majorité sénatoriale travaille depuis des années sur ces questions et que de nombreuses mesures sont régulièrement et voté au cours des différents projets de loi de financement de la. De la sécurité sociale et des différents textes en rapport avec la santé, favoriser le cumul emploi-retraite, simplifier les démarches administratives afin de dégager du temps médical favoriser l'exercice pluri-disciplinaire. Nous sommes régulièrement force de proposition loin de tout dogmatisme est toujours avec le bon sens qui aura qui qui caractérise la Haute assemblée aussi nous continuons de plaider en faveur d'une nouvelle loi santé afin de repenser plus main plus globalement l'accès aux soins dans notre pays en concertation à évêque les différents acteurs de santé, dont bien sûr les médecins pour toutes ces raisons et bien que nous puissions partager à la fois les constats les enjeux de cette proposition de loi le groupe Les Républicains ne votera pas ce texte. Une accumulation de texte n'apparaissant pas pertinente. Faisons confiance aux négociations conventionnelles. Je vous remercie. À l'article 1er, la parole est à monsieur Daniel va te blé pour le groupe les indépendants. Merci madame présidente. Madame la ministre madame le rapporteur mes chèques, mes chers collègues. Je tenais à prendre la parole quelques instants pour évoquer l'amendement que j'ai déposé mais qui a tiré. Irrecevables au titre de l'article 40. Je regrette cette décision. Un maire peut affecter son personnel sur d'autres missions sans aggraver la charge. Il me semble important que ce sujet soit évoqué aujourd'hui. En matière de lutte contre les déserts médicaux, les principaux fantassins sont les élus locaux et en première ligne les mères.-- Ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certains tentent de pallier cette incurie, par des incitations financières conséquentes une commune propose même 50.000 euros de prime à l'installation de nouveaux médecins. Un département voisin du mien. Est engagé dans une aspirine tension le salariat des médecins. 90.000 euros d'investissement. Prise en charge des factures secrétaire médicale et un salaire, ce n'est plus la médecine libérale, même l'État met à disposition des assistants médicaux, depuis la loi Buzyn de 2019. Je voudrais vous parler d'un exemple, l'exemple du maire de confort Philippe monsieur Sonic linkers qui en tribune et que je salue. C'était a pris ses fonctions en 2020 afin de pouvoir maintenir une mission de médical dans sa commune. Il a dit dans l'urgence de proposer la mise à disposition de deux agents communaux afin de réaliser des tâches administratives et de soulager les médecins le de cette charge et cela pendant 8 mois. L'intention est louable. Toutefois, suite à des maladresses dans le processus. Il a été lourdement condamné. Pour détournement de fonds. Triple peine un non dit éligibilité. Une lourde amende et l'inscription au casier judiciaire. L'amendement que je proposais. Proposer de débattre justement pour permettre la mise à disposition d'agents de mairie à des cabinets médicaux ou à des ondes santé, à l'instar de ce qui se pratique pour les du bureau de poste communaux, souvenez-vous en 90 hein enfin de de le maintenir les services postaux dans tous les territoires. Le Parlement a conféré La Poste une mission de contribution à la gym à l'aménagement de ce territoire et pourrait faire de même. Pour les cabinets médicaux et les maisons médicales.

Tout à l'heure, vous avez eu des mots peu agréable à l'égard du président Hollande. En rappelant. Entre guillemets ce que vous estimez être son bilan en la matière. Je n'aurais donc pas de mots et très agréable non plus à à votre égard. En tout cas à l'égard de l'exécutif. Ça a été évoqué par Madame Corinne Imbert, il y a quelques instants, j'avais interrogé monsieur Castex le 18 novembre 2021 pour lui demander quand allez-ce fameux ce fameux décret allait sortir. Pour appliquer la loi de la République, il m'avait répondu, je le cite, au printemps prochain donc printemps prochain en 2022. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur cette incurie gouvernementale manifeste et qui fait que la loi, encore une fois, de la République ne peut pas être appliqué dans de bonnes conditions et pourquoi je vous pose cette question c'est parce que vous-même madame la ministre. Et votre gouvernement dans le cadre de l'article 37 23 du PLFSS. Avait décidé. Cette fameuse année supplémentaire d'études avec il y a un positionnement de ces étudiants en zone. Sous-dense et il y a plusieurs mesures réglementaires nécessaires pour faire appliquer ce texte voté avec le 49.3, ainsi que nous le savons donc je connaissais l'expression populaire, chat échaudé craignant l'eau froide. Je voulais savoir si, finalement, hé bien nous ne sommes pas là dans une forme d'enfumage de la représentation parlementaire au travers donc de mesures réglementaires, que nous allons attendre pendant des mois, des mois, voire même des années votre éclairage Madame Ministre sera très important. Ensuite la parole que je viens de prononcer. Je vous en remercie. La parole est à monsieur Jean-Luc Fichet. Oui madame la présidente. Merci madame la ministre, il y a les déserts médicaux et puis il y a les déserts sur les bancs de la droite qui n'est apparemment pas très intéressée par le sujet, bien que traitant cette question depuis de nombreuses années. J'ai bien compris ce qu'a dit Madame Imbert, tout à l'heure. Le résultat c'est que rien n'avance. Je dirais même que l'on recule puisque aujourd'hui. L'offre de soins dans les territoires diminue se restreint et ça devient un vrai problème, il faut aussi aborder la question du côté des médecins et des professionnels bien évidemment qu'on respecte profondément la profession libérale. Mais pour autant il y a d'autres

Se voient avec aussi des devoirs pour essayer de, de répondre à la demande de la population et puis je voudrais aussi. Traiter la question des des maires ruraux. On ne parle pas ou des maires en général on ne parle pas de et des contraintes que cela va supposer pour eux dans l'investissement qui leur sera nécessaire, et sans aucune visibilité. En fait le problème c'est que depuis des années, on fait des petites mesurettes à défaut d'un vrai projet de santé qui nous avait été promis et depuis 6 ans que vous êtes maintenant au pouvoir. Aucune esquisse dans ce sens-là aucune ambition aucune réponse et donc je voudrais féliciter le rapporteur, madame Héroux pour le travail qu'elle a fait sur un texte qui est justement un texte mesurer un texte équilibré, un texte qui a été travaillé de façon à ce qu'on puisse avancer tranquillement sur ce sujet et vraiment répondre à la question des Français à leurs besoins en matière de santé, je vous remercie. merci madame, la la présidente tout à l'heure Madame la Ministre, vous avez dit que la situation était préoccupante en ce qui concerne l'offre de soins. Moi je crois que le qualificatif est faible, c'est vraiment un euphémisme. La situation n'est pas préoccupant, la situation est dramatique. Elle est dramatique d'ores et déjà pour 87% du territoire national, les chiffres parlent d'eux-mêmes et elle est dramatique pour 6 millions de de nos concitoyens. Et quand on regarde les projections qui sont faites sur une très grande partie des territoires de notre pays. La situation de va que se dégrader au cours des années qui viennent, sur beaucoup de territoires d'ores et déjà quand on regarde le solde entre le nombre de médecins généralistes qui s'installe et le nombre de médecins généralistes qui partent pour des raisons diverses, parfois à la retraite. Parfois ils partent brutalement sur d'autres régions dans des métropoles ou bien sur le littoral ce seul est négatif. D'ores et déjà et donc il va falloir effectivement prendre des mesures fortes des mesures audacieuses ambitieuses et ne plus se contenter de demi-mesure, sinon la situation ne va que se dégrader. Quant aux mesures incitatives. Les mesures incitatives, on peut d'ores et déjà établir un 1er bilan on les connaît les mesures incitatives aujourd'hui on le voit ce qui se passe sur les zones de revitalisation rurale qui représente quand même plus de 15.000 communes dans notre pays et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Les mesures incitatives sur ces ZRR quant effectivement propose 50.000 euros à un nouveau médecin qui vient s'installer une exonération fiscale totale pendant 5 années se sont quand même des mesures incitatives très forte et malgré cela, la situation ne fait que se dégrader et puis je dirai, plus généralement, étant donné cette, cette urgence des urgences parce que c'est cela je crois la préoccupation numéro un de nos concitoyens sur les territoires aujourd'hui derrière cette problématique de l'offre de soins c'est véritablement la question de du crédit de la crédibilité de l'action et de la parole publique qui est dans notre pays, si on n'est pas capable effectivement de donner satisfaction à ce besoin fondamental qui est le respect du droit à la santé, hé bien on ne sera pas crédible globalement.-- Merci la parole est à monsieur Johnny. Merci madame le président, madame le Ministre, mes chers collègues, le. Je voudrais intervenir aussi parce que je considère que j'avais déposé 4 amendements de ont été retenues d'eau était considérée comme recevable. les deux amendements le 1er concernait le forfait urgence patient aujourd'hui que je proposais de supprimer considérant qu'. Il y avait un lien avec le sujet que nous abordons aujourd'hui la désertification médicale parce que sur un certain nombre de territoires et ça a été évoqué plusieurs millions de de de Français n'ont pas de médecin référent donc ils n'ont pas d'autre solution que d'aller aux urgences et se trouve sanctionné parce qu'ils n'ont pas et parce qu'une défaillance du du système de santé qu'ils n'ont pas de médecin référent. Le 2ème élément concernait l'intérim médical là aussi un intérêt médical qui n'est pas satisfaisant qui épuise financièrement nos nos établissements qui ne permet pas de faire fonctionner des. Les équipes de santé de manière cohérente parce que l'engagement d'un intérimaire ne va être le même que que que d'un que d'un agent avec un personnel permanent, et là aussi en limitant la possibilité la durée pendant laquelle on peut exercer son activité médicale par intérim on part on pouvait participer d'une certaine manière, une meilleure répartition dans sur le territoire et également favoriser les installations définitif dans certains établissements. Je vous remercie.-- Madame la ministre, vous avez souhaité prendre la parole. merci madame la présidente. Oui je avais souhaité parce que j'ai été interrogé sur les chiffres. Guillotin qui me poser des questions sur les chiffres tout à l'heure après la discussion générale. pour la rentrée 2022 c'était 303.380, 1000 postes d'internes de médecine générale qui ont été ouverts en 2027, ce sera 4635, soit une augmentation de plus 26%. Mais nous sommes bien en train de travailler aussi sur l'anticipation, puisque l'un d'entre vous a évoqué le sujet de l'anticipation et nous sommes en train de, de monter à un modèle démographique qui prend en compte la pyramide des âges, mais comme ça a été évoqué par bon nombre d'entre vous. Nous ne pouvons plus prendre uniquement à la pyramide des âges comme puisque vous savez très bien que le mode d'exercice a beaucoup changé, que le temps médical et le temps de travail a beaucoup changé et que l'exercice sur lequel nous travaillons c'est-à-dire un transfert de tâches. L'arrivée du numérique aussi. Doit nous permettre de de de constituer un modèle différent mais nous sommes bien dans une phase d'anticipation, pas uniquement d'ailleurs pour la médecine générale et les spécialistes mais aussi pour toutes les professions de santé puisque comme vous le savez, nous manquons aussi d'aide-soignantes et d'infirmières, c'est un des enjeux de de du groupe de travail dans des CNR nationaux qui seront lancés très prochainement. Je voulais dire que j'étais en Aveyron lundi est. Ce que vous avez décrit, Monsieur le Sénateur ne corrobore que l'idée que le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la, la charge qui s'appelle organisation territoriale. Ce que vous avez décrit, montre bien que la nouvelle la méthode souhaitée par le président de la République et la Première ministre c'est partir des territoires et travailler avec les territoires pour apporter des réponses. C'est bien l'enjeu qui est le nôtre, c'est bien ce changement de méthode que nous soyons que nous voulons porter. Et je peux vous dire que je fais beaucoup de déplacement en ce moment et que notamment à travers les CNR qui sont en train de se dérouler, qui sont en train de se terminer. Nous voyons bien que des propositions émanent de tous les territoires qu'elles peuvent être adapté à d'autres. Nous allons accompagner les territoires qui font des propositions rapidement et nous le souhaitons le faire, mais nous mettrons aussi à disposition dans cette fameuse grande boîte à outils d'autres territoires des solutions innovantes et intéressantes. Qui proviennent d'autres territoires. L'idée, c'est bien de partir des territoires pour remonter vers la haut, et de plus décidé de façon unilatérale. D'une décision qui s'appliqueraient dans tous les territoires. Je suis intimement convaincu que ce que j'ai vu à Saint-Georges de Luzon sont ne pourrait pas être appliquée en Île-de-France qui est le plus grand désert médical de France, je le rappelle. Monsieur le sénateur Wattebled votre proposition et votre amendement qui a été rejeté. Nous sommes en train de l'expertiser avec la une société parce que nous pensons que, effectivement, peut-être il serait possible au maire de mettre à disposition du personnel dans les maisons médicales. C'est bien l'enjeu de l'expertise que nous, nous avons lancé avec la une c'était. Expertisée ne veut pas dire. Mais nous avons lancé l'expertise. Je vous rappelle pour ceux qui. N'ont dit qu'il y avait pas eu de proposition de loi de projets de loi fait sur la santé ma santé 2022 il me semble bien qu'c'était une. Un projet de loi de santé et puis, la situation est tellement préoccupante que je ne cesse de dire que nous sommes dans le mur. Puisque 87% de la France est est un désert médical. Et nous sommes aussi intimement convaincu que puisque nous sommes dans le mur c'est bien ensemble à la fois les élus locaux, les professionnels de santé les usagers qu'il ne faut pas oublier aussi dans les propositions à faire, que nous allons. Trouver les réponses à la fois avec la coordination entre les professionnels de santé. La coopération entre les élus, les professionnels et les usagers et non pas de la coercition.-- Bien nous allons passer à l'examen des amendements avec 2 amendements qui font l'objet d'une mission commune, Monsieur Chassaing le le 8 et le sept, vous les défendez l'un après l'autre où ils sont défendus par votre intervention, je vous voyais les. C'est à vous.

alors si vous voulez. Cependant, dans sa rédaction actuelle. Le texte prévoit que cette année soit fait. Tu es auprès de maître de stage universitaires Dans les territoires ruraux, certains médecins qui ont beaucoup de clientèle mais n'auront peut-être pas les moyens ou le temps d'aller se former en comme maître de stage. C'est pour ça que je proposais que le stage dans sa dernière année, puisse être réalisée. Six mois avec un maître de stage et 6 mois avec un médecin traitant. Qui serait un médecin référent. Je dois quand même dire que la dixième année d'études médicales, c'est-à-dire après 3 ans d'internat. On met à nouveau une 4ème année d'études. Ben le, le, le médecin qui sera un médecin, un médecin junior. Pourrait déjà dans cette 4ème année c'est n'existait pas faire des remplacements. Donc moi ce que je propose, c'est effectivement si mois avec un maître de stage et la possibilité les 6 derniers mois. d'aller avec un médecin traitant qui serait le médecin référent et ça permettrait de, de le, de soulager ce médecin est peut-être lui permettre aussi de s'associer dans un 2ème temps merci le le 2ème amendement si vous voulez, c'est un autre amendement qui est dans le même sens, c'est un an avec un médecin traitant mais je pense que je soutiens plutôt cet amendement que je viens de détailler, merci. Merci. Quel est l'avis de la rapporteure sur ces amendements.-- Merci madame la présidente.-- Sénateur Jacinthe ces deux amendements donc. Auront un avis défavorable en effet le il nous apparaît que le statut de maître de stage universitaire. Est important. Il suppose une formation préalable à l'agrément. Il permet d'assurer la qualité de l'encadrement des jeunes médecins en année de professionnalisation. Le nombre de maître de stage universitaire a beaucoup pour augmenter ces dernières années. Et il continue de. Croître grâce aux efforts conjugués des universitaires et des collectivités. De plus il ne paraît pas souhaitable de scinder. L'année de professionnalisation en 2 semestres auprès de de praticiens distincts, un exercice long préférable pour favoriser tant l'autonomie du jeune médecin, que son installation dans le territoire et donc, en conséquence la commission a émis un avis défavorable à ces deux amendements. Quel est l'avis d'un du gouvernement.-- Le gouvernement est particulièrement vigilants à la qualité de l'encadrement pédagogique des futurs professionnels de santé pour les mêmes raisons évoquées par la présidente. Par la rapporteure. Le Gouvernement émet un avis défavorable à ces deux amendements.-- Merci je vais donc. Monsieur Jomier.-- Merci madame la présidente. Alors j'ai effectivement moi je soutiendrai pas non plus l'amendement Daniel Chassain parce que je pense qu'il faut être. Respectueux. Enfin je sais que Daniel les mais il faut être, faire attention au message qu'on envoie aux jeunes médecins et ils nous demandent que ceux-ci on leur. leur. Demande de faire une année de plus, il y a un encadrement qui soit un encadrement par un maître de stage universitaires et d'ailleurs moi j'appelle à ce que dans toutes les dispositions qu'on adopte on prenne garde à ne pas brutaliser les jeunes médecins. Les internes sont en souffrance, ils nous le disent sans cesse. Ça ne se passe pas bien dans les hôpitaux de façon récurrente parce qu'ils sont soumis à des rythmes qui sont très élevées et on les rémunère pour remplir une fonction essentielle de façon qui n'est pas satisfaisante. Or dans cette année supplémentaire, c'est le problème du texte du gouvernement comme je le dis, c'était le problème de la PPL que que vous avez adopté sur proposition de Bruno Retailleau en disant que c'est une 4ème année d'internat, ça fait forcément référence à ce qui est la rémunération d'un interne et en disant que ce n'est pas une année d'internat, mais une année de professionnalisation. Ça ouvre un autre statut et donc une rémunération plus élevée et c'est juste et c'est pour ça que je défends cet article 1er et comme j'ai encore quelques secondes. Je voudrais dire à Madame la Ministre hein que le rôle des maires c'est pas par l'expertise, un amendement qui se règlent, c'est en modifiant la loi sur les compétences et les occasions n'ont pas manqué notamment lors de la loi 3DS et à chaque fois, le gouvernement a refusé d'étendre la compétence des maires en la matière. Si les mères avaient la compétence, hé bien il n'aurait pas les problèmes qui ont été rappelés par notre collègue et donc moi j'appelle le gouvernement plutôt à légiférer pour qu'on modifie qu'on reconnaisse le rôle des collectivités territoriales sur la santé et pour terminer en quelques secondes la politique de l'offre qui était celle de la restriction du nombre de soignants formés vous la poursuivez largement avec un Ondam de soins de ville égal à la moitié de l'inflation et un égal un Ondam hospitalier inférieure à l'inflation.

ne va pas être rémunérés comme des internes, c'est pour ça que je proposais. 10 consultations par jour sur 5000 euros par mois. Mais. Si vous voulez pourquoi j'ai proposé cet amendement, c'est parce que si on veut être efficace dans le milieu rural où on a des médecins qui vont être peut-être à 60 65 ans qui ne vont pas vouloir être maître de stage qui ont une énorme clientèle et qui dedans et qui dans cette conception pourtant en pourtant en ayant un étudiant qui en dixième année qui a fait trois ans d'internat, alors qu'avant je rappelle qu'on faisait des remplacements. En étant interne. Donc je trouve quand même que c'est excessif et que on pourrait permettre. Peut-être les 6 derniers mois, de permettre à un médecin traitant qui serait médecin référent d'avoir un interne qui vient l'aider et qui serait en quelque sorte un médecin remplaçant mais qui pourrait être. Le médecin référent là le le le médecin junior rencontre un problème ou avoir un avis pour aiguiller au mieux sont malades. Voilà et je pense que dans la vraie vie c'est ça serait très bien, effectivement on me dit que c'est mal et donc je vais retirer mes amendements.-- Merci, nous allons donc. Maintenant passer à l'amendement de madame Pumerole.-- Madame Pumerole. Oui merci madame la présidente. Nous avons présenté l'idée qu'il fallait que ce soit au niveau du une commission départementale. Que l'on puisse avoir, donc l'accompagnement et l'aide à l'installation. D'abord l'aide je dirais à. À la réalisation de l'emmener de professionnalisation dans les territoires sous ôter. Mais nous avions mis dans la première version que dans la commission serait présente des membres de l'AMF. Or il existe plusieurs associations de de mer, il existe aussi la saucisse seconde maires ruraux et donc il me semblait plus simple de corriger, juste sur le plan rédactionnel. Le fait qu'on puisse mettre des mères à la place donc de l'Association des maires de France.-- quel est l'avis de la commission sur cet amendement madame la rapporteure.-- Pardon. En fait la commission ayant rejeté le texte il a émis un avis défavorable à cet amendement à titre bien personnel bien sûr, je crois qu'il serait souhaitable de reprise de remplacer effectivement ce représentant des communes du département. Que les qu'un représentant des communes du département participent à ces commissions départementales. Les collectivités en effet joue déjà un rôle. Important dans l'accueil des étudiants, stagiaires, et plus largement dans les politiques d'attractivité visant à favoriser l'installation des médecins l'amendement donc se borne à substituer un représentant de l'AMF qui était initialement prévu par le texte par un représentant des communes parce qu'il y a parfois des maires investi qui sont membres de par exemple à l'Association des maires ruraux de France et ces maires pourraient participer à cette commission départementale. Donc nous voulons être le plus ouvert possible.-- Très bien. Madame la Ministre quel est votre avis sur cet amendement. Vous proposez de prévoir que la commission d'affectation et d'accompagnement à l'exercice de l'année de profit délégation qui chargé de fixer la liste départementale et l'université, c'est un médecin généraliste, qu'on prenne un représentant des communes du département au lieu d'un représentant départemental de l'Association des maires de France. Or, à mon sens il n'y a pas de différence entre ce que vous proposez et ce qui est écrit dans le texte initial. L'Association des maires de France représente chaque commune, du département, son représentant départemental et donc en mesure de représenter les communes du département. De plus, afin d'organiser la mise en oeuvre de la 4ème année d'internat de médecine générale. Une mission a été confiée par le gouvernement à 4 personnalités qualifiées. Cette mission a d'ailleurs auditionné les représentants des principales associations représentatives des collectivités territoriales pour toutes ces raisons, cet amendement étant déjà satisfait. Je vous propose de le retirer sinon j'y serais défavorable. je vais mettre aux voix cet amendement qui a un double avis défavorable qui est pour.-- Qui est contre. Il est adopté.-- Alors sur l'article 1er, nous allons procéder à un scrutin public, à la demande du groupe les républicains. Madame Casabonne appelle un huissier. Le scrutin est ouvert.

pour 97 contre 196, le Sénat n'a pas adopté l'article 1. Nous passons à l'article 2 et un nouveau scrutin public.-- Le scrutin est ouvert.

plus personne ne demande à voter Le scrutin est clos. Votants 317 exprimés, 297 pour 99 contre 198. N'a, n'a pas adopté.-- Nous passons donc maintenant à l'article 3 qui fait l'objet d'une nouvelle demande de scrutin public.-- Le scrutin est ouvert.

Nous passons maintenant à l'article IV. Même procédure même scrutin, scrutin public. Le scrutin est ouvert. c'est qu'il y a des problèmes d'écran. Depuis ce matin et les services de la DSI sont. S'en occupe et cherche à. Vous offrir le meilleur écran.

Plus personne m'en noté le scrutin est donc clos. Votants 318 exprimes, 315 pour 120 contre 195 après l'article IV.

Madame la présidente à la unissent mes chers collègues. L'amendement 14. Et et le suivant. Il s'agit de faciliter ou de renforcer la fesse, l'accès aux soins. Aujourd'hui ils constituent une urgence dans les territoires. Les conséquences de cette difficulté d'accéder aux soins et dramatique. On a sur des territoires des fréquentations médical des consultations deux fois moindre, et même plus que la moyenne nationale. Ce qui est c'est un n'est pas la seule raison bien sûr mais génère une espérance de vie qui qui est plus faible. Jusqu'à 4 à 5 ans de moins sur Saint a été Édouard en France si on ajoute à cette inégalité territoriale inégalités soit sociale les inégalités en termes d'espérance de vie peuvent atteint 13 années ce qui est quand même une inégalité inacceptable. Il nous faut aujourd'hui Gerry la paix la pénurie. La situation aujourd'hui dans le territoire et ça a été dit, génère une insécurité totale de la part de nos populations, en particulier dans les territoires où la population est vieillissante, donc avec un besoin de Sion soins que vous le connaissez et en particulier dans les territoires ruraux.-- Il s'agit de faire une proposition qui n'est pas contre les les les étudiants pas contre les médecins qui viennent d'être formés, il s'agit pas d'ailleurs d'une coercition, mais plutôt d'une oeuvre de régulation. Soyons attentifs aux mots qui sont. les mesures incitatives ça été évoqué avant moi. Aujourd'hui, elles sont nombreuses et et très avantageuse ne sont pas suffisantes, il faut aller au-delà. D'où l'ma proposition. Pour les étudiants qui sont formés et qui souhaitent exercer leur médecine leur activité dans une zone sur-dotée, on leur demande et de de de s'installer temporairement temporairement dans une zone normale pendant 12 mois. À faire sur 3 ans s'il le souhaite pour prendre en compte leur problématique familiale, ils sont dans des zones urbaines et ils doivent pouvoir éventuellement. Et continuer à avoir une vie de famille, mais faire une heure ou une heure et demie par an j'ai j'ai je vais présenter les 2 rapports. Les 2 amendements. Madame la présidente. Ce qui peut expliquer que non que je prenne un petit peu de temps et donc leur proposer assez à ses étudiants formés d'exercer leur destine pendant 12 mois sur une période de 3 ans, ils le font soit en une seule fois, soit sur la durée, en venant faire des présences médicale une semaine eu un jour un jour et demi par par semaine sur cette période, ce qui permet de, d'avoir une passion telle et et de la suivre et de pouvoir effectivement exercer également en en dans les zones métropolitaines urbaines ou urbaines denses et bien évidemment pouvoir avoir la vie de famille et notamment prendre en compte la problématique du conjoint. Ces 12 mois sont réduits à six mois dans les zones sous-dotées c'est-à-dire les ce qu'on appelle les déserts médicaux ne va des étudiants formés qui ne souhaite pas exercer la médecine devant des patients qui soient travaillent dans des laboratoires soit dans assurance sur leur demande de faire six mois sur un territoire sous-doté à la sortie de leur de leur formation avant d'exercer leur activité professionnelle. Et puis, permettez-moi d'ajouter une nuance. On a, on a dit qu'aujourd'hui selon des modalités de calcul qu'on peine à à maîtriser qui à mon avis mériterait d'être révisé. On considère que, aujourd'hui en France il y a que 13% de de notre territoire qui est considéré comme étant en zones surdotées. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, on a une pénurie. On peut calculer une moyenne de présence médicale par rapport à la population. Est en zones surdotées tout territoire qui a une présence médicale supérieure à la moyenne est en zone sous-dotée tout territoire qui a une présence médicale inférieur à la moyenne nationale. Il va falloir travailler par rapport à ça parce qu'il y a une pénurie effectivement qui va durer encore au moins une dizaine d'années, il va falloir apporter des réponses de long terme et sortir des approches théoriques de ce qui constitue un encadrement satisfaisant de la population sur le plan médical, je vous remercie.

L'amendement propose un mécanisme plus contraignant que le conventionnement proposée à l'article IV. En outre il n'évite pas la surconcentration des médecins en zones surdotées ne permettrait donc pas une répartition équilibrée des professionnels sur le territoire. La commission a a donc émis un avis défavorable, donc c'est un, une demande de retrait ou un avis défavorable. Concernant l'amendement numéro 15 hein. On comprend bien l'intention de résorber les pénurie, la pénurie de de médecins généralistes dans les zones en difficulté. Pour autant. La méthode employée ne me semble pas tout à fait convaincante l'amendement près supposerait que la médecine générale puisse s'exercer entre guillemets entre guillemets au pied levé. Or il s'agit bien d'une spécialité en soi à laquelle les internes en médecine générale sont formés. Il ne serait pas opportun de créer des médecins généralistes contre leur gré ou sans formation spécifique adapté. À vie donc défavorable de la commission, madame la Ministre. Merci madame la présidente. Donc un avis défavorable. Vous proposez de conditionner le conventionnement en zones surdotées un exercice préalable équivalent à au moins 12 mois en ETP sur 3 ans en zone que vous qualifiez de normal la contrainte à la Stala Sion n'est pas la solution.-- Introduire une coercition l'installation conduirait inéluctablement un grand nombre de médecins a retardé leur installation ou à s'orienter vers des solutions de contournement. Ceux-ci risqueraient d'aggraver encore les problèmes d'accès aux soins. Les résultats d'ailleurs très mitigé des dispositifs de conventionnement coercitif mise en oeuvre en Allemagne par exemple démontre. Bien les Bien les limites de ce type de mesure. Par ailleurs, il est difficile d'identifier des zones sur-denses pour les médecins, en particulier les médecins généralistes car les difficultés démographiques affectent aujourd'hui la quasi-totalité du territoire national, 87% de la France est un désert médical. En outre, dans les zones moins sous-dotés les projections démographiques indiquent souvent un nombre important de départs alors traite de médecins dans les 5 prochaines années. Pour ces raisons je suis défavorable à cet amendement concernant l'amendement 15 un avis défavorable. Si vous proposer de mettre en place une obligation générale d'exercice en médecine générale pour l'ensemble des nouveaux diplômés qui n'exercerait pas devant les patients une telle généralisation reviendrait à nier la spécificité de la médecine générale toute internes de médecine n'est pas directement au contact d'un patient au cours de sa formation initiale, c'est le cas des étudiants en santé publique leur formation vise à former des médecins à une approche collective, des problèmes de santé capable d'apporter une expertise médicale aux questions posées en termes de santé des populations et de contribuer à l'argumentation des politiques sanitaires par ailleurs nous n'entendons pas contraindre la liberté d'installation pour ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Madame mon Jean. Explications de vote.

Mais enfin quand même l'adresse hein qui est un organisme quand même sérieux et scientifique montre bien qu'il y a une gradation quand même dans la densité médicale et elle dit notamment que je l'ai dit dans mon intervention générale que 30% est en zone d'intervention prioritaire, là on a vraiment une priorité. Ça c'est dans le terme même de zones d'intervention prioritaire et ensuite les zones quand même un peu mieux dotées. Il y a quand même les. Les zones le deuxième la deuxième couche les zones d'actions complémentaires qui sont pour un peu plus de 40%, c'est-à-dire qu'on a 75%. Du territoire qui est, qui peut être. Définie comme des zones soit prioritaire soit nécessitant des des actions complémentaires. Alors je dirais que par complément. Bon moi je mettrais pas la moyenne mais qui par complément effectivement vous avez 25%.

politique publique. C'est le titre d'ailleurs de la PPL en termes d'équité territoriale, donc arrêtons de de de de mettre ça sous un, un terme un peu général. C'est partout pareil et caetera, non c'est plus ou moins profond. Il y a dégradation et ses gradation s'approfondissent, donc il faut agir pour plus d'équité et c'est le titre de cette PPL.-- Très bien je suis saisie sur cet amendement 14 une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains.-- Le scrutin va être annoncé. Il est annoncé, il est ouvert.

Plus personne ne m'en a voté le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 276 pour 7 contre 269.--

Alors si vous voulez moi pour moi. L'article 5 pose le problème d'une égalité de traitement entre les médecins libéraux et les médecins salariés en matière d'aide publique. Donc compte tenu des particularités de chacun des modes d'exercice cette égalité n'est pas juste. Les médecins libéraux. Prennent des risques, ils vont s'installer dans une maison de santé pluridisciplinaire ils vont gérer, d'abord ils vont payer leur, leur secrétaire ils vont payer un loyer donc. À la commune ou la communauté de communes qui a qui a fait la maison de santé. Et ils vont gérer en association. La maison de santé. vous voulez, il ne s'agit pas de bien sûr de hiérarchie des modes d'exercice mais seulement de reconnaître que les statuts sont différents et le volume de travail des médecins libéraux permet de protéger davantage de soins que les médecins salariés. Donc si le salariat répond effectivement aux aspirations de nos médecins ça c'est. Je pense possible à l'hôpital où il y a de nombreux médecins notamment aux urgences où il y a des heures précises. Mais si vous voulez. La médecine libérale est aujourd'hui, je pense en mesure de résoudre les difficultés d'âge. D'accès aux soins, tout particulièrement en zone rurale. Donc il faut encourager ces médecins qui prennent quand même des des risques pour s'installer et qui vont bien sûr pour. Avoir. De. L'accès aux soins de des personnes pour les soins non programmés. Ben ils vont faire des heures plus importante et je pense que il faut absolument les encourager. Et donc c'est pour ça que je ne suis contre l'article 5.-- Quel est l'avis de la commission.-- pouvant fonder une distinction dans l'octroi des aides. Je voulais juste prendre un exemple, les contrats incitatif prévoit par exemple des montant et des modalités différentes pour les médecins pour un praticien travaillant à temps plein en zones sous-dotées. L'aide est ainsi de 50.000 euros pour un exercice en libéral compte contre 30.000 euros pour le premier équivalents temps plein au sein d'un centre de santé. Donc je pense que le risque pour le les porteurs du projet de Centre de santé justifie aussi le la même aide. À titre personnel, donc je considère que l'exercice salarié de la médecine contribue aux soins de 1er recours au même titre que l'exercice libéral. Il est donc normal que les aides ne soient pas discriminante et qu'elles incitent équitablement atteint à travailler dans les zones sous-denses.-- Un avis favorable à un des enjeux aujourd'hui hé bien de répondre aux aspirations des jeunes médecins qui peuvent être différentes dans les choix du d'exercice soit salariat soit libéral. Je souscris à votre argument selon lequel il n'y a pas de hiérarchisation des modes d'exercice. À noter que des dispositions conventionnelles régis par le code de la sécurité sociale prévoit bien une transposition des dispositions de la convention nationale médicale au centre de santé. Le contrat d'aide à l'installation comme vous venez de le dire madame la sénatrice, des centres de santé médicaux polyvalent. Et transposition identique et du contrat c'est AIM accessible pour les médecins s'installant en libéral ainsi sous condition de maintenir le Centre de santé pendant 5 ans dans la zone sous-dotée et de participer à la PDSA, le Centre de santé peut bénéficier de 30.000

cette disposition vise justement à favoriser un choix libre avec des conditions. D'installation et des avantages et des jets qui soit neutre que l'on exerce son activité en activité libérale ou que l'on l'exerce comme salariés d'un centre de santé il me semble que cohérent effectivement de faire en sorte qu'il y a une forme de neutralité dans l'accompagnement, l'installation des médecins c'est comme ça effectivement qu'on permet un choix libre aux jeunes médecins pour s'installer dans les territoires en manque de professionnels de santé, en choisissant ce qui leur convient le mieux au regard à la fois de leur de leur envies professionnelles et de leur choix personnel. Madame Pumerole. Oui merci madame. La présidente lorsque nous avons rédigé cet article. Nous avons pensé effectivement à ce que vient d'évoquer, mon collègue Patrice Joly à la liberté d'installation. C'est un principe important et effectivement il nous semblait anormal qui une discrimination entre l'exercice libéral et l'exercice en cendres santé il n'est pas question d'opposer l'exercice libéral et de l'exercice en cendres santé ils sont complémentaires. Mais on doit pouvoir permettre à chaque jeune médecin de choisir l'exercice qui lui paraît le plus intéressant pour lui, comme vient de le dire mon collègue joli en fonction de ses. Envies ou ses goûts. Particuliers et donc l'idée d'avoir une discrimination et qui est importante puisque, en centre-santé ça vient d'être rappelé encore par Madame le Ministre c'est 30.000. pour un équivalent temps plein, ça n'est plus que 20.000 pour le second. On y a droit que pour 3 médecins. Installés dans le centre de santé alors que dans une MSP dans une maison de santé pluri-professionnelles qui serait. Donc en zone sous sous douter pareil c'est 50.000 euros et quel que soit le nombre de médecins qui seraient installés donc le, le différentiel est quand même suffisamment important pour qu'on puisse. Le souligner et proposé, il soit supprimé avant qu'il ait une véritable liberté de choix pour le aux jeunes étudiants. Dans le mode d'exercice, ce qu'ils veulent exercer. Merci madame Cohen.

en en salariat ensemble de santé me, me paraît extrêmement important mais je pense aussi, mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est quand même méconnaître l'activité des centres de santé aujourd'hui dans au niveau des centres de santé, outre le fait qu'il y a une appétence des jeunes médecins à y travailler parce qu'ils ont envie de travailler en équipe, ils ont envie de travailler. Aussi en en tant que salarié pour être déchargé. De tout ce qui est administratif, etc mais il y a aussi cette volonté très forte. Je le redis, de travailler en équipe, sans. Dépassement d'honoraires et c'est un peu sur le même mode d'exercice d'ailleurs que l'hôpital et ne pas voir cette appétence ce désir et cetera c'est ne pas encourager justement les jeunes médecins à pouvoir s'installer là où ils l'entendent et donc alors que l'on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés à. Recruter des médecins d'ailleurs, y compris dans les centres dans santé, c'est difficile, je pense que on continue à mettre du des bâtons dans les roues avec une idée je dirais idéalisée de l'exercice libéral. Moi je pense qu'il ne faut pas de discrimination, qu'il faut encourager les modes d'exercice seuls en cabinet en en maison de santé ou en centre de santé, pour permettre vraiment un vrai maillage dans nos territoires, qui en ont tous besoin et je pense que ces discriminations, elles doivent être tout à fait gommer parce que nous, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence absolue.

Mais comme dire que un élément de différenciation, c'est qui concentrent qui consentent des sacrifices ne consentiraient donc pas le médecin salarié voir les médecins hospitaliers. Je trouve que vraiment là. Ce et sorte des sacrifices. Je trouve ça un peu choquant mais je reviens sur le fait. Que vous dites, le volume du travail des médecins libéraux et et supérieur. C'est un fait et que. Vous en vous entraîner la conclusion que seule la médecine libérale est aujourd'hui en mesure de résoudre les difficultés d'accès aux soins. Retour au réel, quand même, je renvoie au titre d'ailleurs de cette PPL on constate quand même que en plus la médecine libérale que peut être que d'autres n'assure spontanément l'équité territoriale elle laisse prospérer des zones de plus en plus désertés par les médecins libéraux ou elle fait l'offre en secteur hein donc. Moi je je je renvoie à d'autres expériences. Répondant à une aspiration quand même de réduire son temps de travail et ce quels que soient les statuts certains territoires n'hésite pas faciliter l'ouverture de centres de santé justement comme le département par exemple de Saone-et-Loire qui qui est parvenu à attirer 70 médecins de statut salarié et rien n'empêche et soignants et d'ailleurs c'est le cas de travailler en heures supplémentaires et en conséquence de pratiquer autant de soin que les médecins libéraux notamment les nouveaux qui ne travaille pas comme avant. Donc il ne faut pas parler des des anciens mes médecins libéraux par rapport au nouvel exercice. Salarié donc cette démarche issus des territoires montre bien que la solution passe aussi par les médecins salariés libéraux ou salariés. La spécialité de médecine générale relève des mêmes motivations et nous deux doit faire l'objet donc des mêmes attention voilà. Et si notre objectif est de lutter sérieusement contre les déserts médicaux. Toutes les solutions doivent être envisagées en octroyant le même niveau d'aide. Pour si Madame je passe la parole à Monsieur Chassaing. La présidente, mes chers collègues. Moi je suis pas du tout compte, les médecins salariés. Je suis pour la liberté d'installation dans mon amendement je souhaite favoriser l'installation des médecins libéraux. Ben c'est tout je je pense que un médecin libéral qui va s'installer dans une maison de santé. Va ne pas compter ses heures. Mais je, je ne dis pas que je retire le mot sacrifice, je retire le mot sacrifice. Je dis que pour un médecin qui va s'installer dans une maison, il ne va pas obligatoirement compter ses heures et et et il va en plus s'occuper de la gestion de la coordination de l'association avec les paramédicaux et je pense qu'il faut encourager les médecins qui veulent s'investir. Dans les maisons de santé et bien sûr les centres de santé, ça peut être en ville le le les départements peuvent créer des centres de santé avec des, des médecins

dans mon amendement vous vous souhaitez que tout le monde et le le la même dotation publique que ce soit en libérale ou un salarié, moi je dis non je voudrais conserver ce qui c'est ce qui existe actuellement. Ce que propose le gouvernement, c'est-à-dire favoriser l'installation de médecins libéraux, c'est tout.--

sur des territoires Soudan c'est il y a des aides incitatives. Il y a également des aides au centre de santé il faut pas dire que les centres de santé sont pas aidé en tout cas nous en région, on a également font l'ARS est présent quand il y a des centres de santé et des Centres mutualistes qui se monte, mais on ne peut pas dire enfin on donne.

pour autant antinomique. Donc moi je, je voterai pour l'amendement Daniel. Monsieur Jomier.-- Merci madame la présidente, moi je partage la préoccupation de mes collègues qui souhaite que. et c'était le sens de de l'amendement. J'ai j'ai bien compris de de Patrice Joly qu'on traite à équidistance et de la même façon, ceux qui souhaitent tel ou tel mode d'exercice c'est aussi un choix de vie. Le mode d'exercice et il faut le respecter. Moi je voudrais attirer l'attention hein sur le fait que la question de ces aides. Doit être discuté, a commencé à être discuté dans le cadre des négociations, la nouvelle convention qui sont en cours et que tout ça doit être revue. Parce que ça a été dit, les aides sont pas inefficace totalement mais enfin il y a un montant qui est attribué. Qui ne produit pas on va dire, la meilleure efficience deuxièmement est important le destinataire de l'aide. Ce n'est pas la même chose que ce soit directement le professionnel de santé ou que ce soit la structure dans laquelle il existe le professionnel de santé, ce qui m'amène au 3ème point c'est que j'attire aussi l'attention du gouvernement sur la nécessité de prêter vraiment. De prendre des mesures car se développent des centres de santé qui n'ont rien de sympathique et qui pratique de l'optimisation de ces aides, notamment à côté d'autres types d'optimisation de grands groupes privés qui voilà oui bah low cost. On connaît ça et ils sont champions pour justement collecter ces aides les optimiser et développer leurs bénéfices à l'arrivée et ça ne se fait pas, ça ne se fait pas au bénéfice de la qualité des soins et de la qualité de l'exercice des professionnels de santé concernés. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut affronter, on peut accuser l'amendement de ne pas être parfait sur cette question amendement est parfait mais elle a le mérite de poser le problème.--

et il faut le prendre en compte. Vous nous expliquez. Que les médecins en profession libérale sont épuisés, ils ont des charges très lourdes et cetera et ils sont pas assez payés et vous nous expliquez aussi que ils pourraient continuer bien au-delà de la retraite. Plusieurs années à exercer dans ces conditions difficiles parce que là ils sont plus épuisé du tout mais quand on vous dit, oh il y a il y a une alternative. Il y a une proposition qui permet de diversifier l'offre, à travers des centres de santé, mais il faut pour cela que les aides soient équitables. Vous nous dites. Ah ben non c'est pas la même chose ne Centre de santé. Il a d'autres moyens. Il nécessite pas autant de de financement que la l'installation, professions libérales, moi je trouve qu'il y a. Un certain nombre d'explications qui s'opposent dans ce que vous nous dites et qui rend l'exercice vraiment très difficile, je vous remercie.-- Bien je vais mettre aux voix cet amendement six. Monsieur Chassaing voulait retirer votre amendement. Non mais dans ce cas je ne peux pas vous redonner la parole vous avez déjà présenté votre amendement FN, explication de Monsieur blé peut faire une explication de vote.-- Juste pour un scrutin public c'est tout.--

Ça pourrait équivaloir OK donc on n'a pas de demande de scrutin vous la retirer très bien donc je mets aux voix cet amendement qui a reçu un doublé défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Voilà, il n'est pas adopté. Nous avons ensuite un scrutin public sur l'article 5 1. Est ce qu'on pourrait considérer que c'est le même vote que sur les articles précédents.-- on voit au scrutin public. Le scrutin est ouvert.

Plus personne lambda voté le scrutin est clos. Votants 320 exprimés, 308 pour 95. 15 contre 213, le Sénat n'est pas adopté l'article 5. Nous allons passer l'article 6 je vous rappelle pas à voter n'était pas adopté, il n'y aurait pas lieu à voter sur l'ensemble du texte et que donc, c'est maintenant que devrait se faire. Des explications de vote y en arrêt. Madame Préville s'est inscrite pour une explication de vote. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, puisqu'il en est ainsi et qu'il ne restera rien de ce texte. Je souhaite intervenir pour à tout le moins dire ma déception. Effectivement, tout le monde l'a dit, nous sommes face à une situation désastreuse jamais connu, et ce depuis longtemps, je ne sais pas combien de temps il faudrait revenir pour avoir ces difficultés d'accès aux soins. Chaque Français est confrontée à ces difficultés de ne pouvoir avoir un accès normal aux soins et particulièrement à des spécialistes je vous parle en tant qu'élu d'un territoire rural et je vous l'ai dit, les Français ne comprennent pas ce qui est en train de se passer ne comprennent pas qu'on agisse pas et ne comprennent pas qu'il y ait tant de difficultés à résoudre cette situation. Je souhaitais également vous interroger sur ce qui est fait pour améliorer cette situation et notamment vous demander s'il y a assez de moyens qui sont déployés dans les facultés de médecine sur le nombre de places ouvertes de salle d'amphi de laboratoire est ce que l'on permet à tout étudiants désirant devenir médecin de pouvoir étudier. Est-ce que l'accès aux études de médecine a été facilitée. Combien d'enfants d'agriculteurs et d'ouvriers peuvent devenir médecin actuellement est-ce que cela a changé depuis ces dernières années ou pas. Je souhaitais aussi vous interpeller sur le fait de, d'une, de, de ce que d'une des choses que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que c'était au territoire de s'organiser. Les élus consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour bricoler des solutions sans savoir où cela les mènera et si leurs solutions seront efficaces et dire tout simplement que les territoires doivent s'organiser, à mon sens, ce n'est pas acceptable. Voilà ce que je souhaitais vous dire et pour terminer de parler puisque beaucoup a été parler de coercition. Je voudrais

Le travail que nous avions effectué au niveau du du groupe socialiste. C'est un travail d'auditions et de dos à répétition. Nous nous sommes retrouvés souvent dans les auditions, et j'ai pensé que nous aurions l'occasion là de pouvoir discuter ensemble de ce problème majeur, ça vient d'être redit. Qui touche dans l'autre, et vous le savez bien puisque la chambre haute et la représentante des collectivités territoriales qui inquiète énormément nos élus locaux et qui intéresse et qui inquiète évidemment nos concitoyens. Par la technique du scrutin public systématique à chaque article ça vous a permis d'être à un ou deux présents.-- Vous les sénateurs et sénatrices donc 2 des républicains et de emporter bien sûr le vote puisque avec le scrutin public votre présence n'est pas obligatoire et. La présence ne serait rien. Le fait que nous n'avons pas pu discuter. Alors moi je voudrais reprendre Madame la Ministre, vous nous avez dit que nous étions très contraignant. Sur l'article 1, la contrainte n'est pas plus importante que celle que vous avez mise à la suite de la PPL Retailleau dans votre article 23 du PLFSS. Parce que vous imposez un stage. Rémunéré comme un stage interne alors que nous parlons de négociations et de négociations avec des rémunérations qui sont. J'allais dire, donc ne. Avec des internes dans notre article de nous parlons de l'exercice coordonné. Je vous rappelle que l'Ordre des médecins c'est pour Londres, c'est l'Ordre national des médecins s'est prononcé il y a peu pour Me cette obligation dès 2026 et donc. Nous on nous ne sommes pas plus coercitif que l'Ordre des médecins. L'exercice coordonné et favoriser depuis 4 5 ans, malheureusement on attend on attend on a aujourd'hui à peine 220 ESP qui sont montées en France, ce qui fait vraiment extrêmement peu sur l'article 3 sur la sur Nous parlions pas de garde individuelle. Nous demandons à ce qu'on redéfinisse les zones en concertation sur les territoires avec les ARS et avec les CPTS pour définir des zones de garde qui soit intéressante pour tout le monde, enfin sur l'article.

Je n'ai pas d'autres demandes d'explications de vote. Si Monsieur Effectivement tous les médecins qui sont tous les sénateurs qui sont dans dans des territoires ruraux ont beaucoup de soucis et. Malheureusement. le numerus clausus a bien sûr été enlevée, mais il a été enlevé, bien trop tard et on on a plusieurs années. Je peut-être jusqu'en 2030 à avoir beaucoup de problèmes donc ça. Bien sûr. ça ne va pas se résoudre comme ça du jour au lendemain. Alors dans cette proposition de loi. Effectivement, moi je suis d'accord que. Plutôt d'accord sur pas mal d'articles parce que. On est plus dans l'internat, si vous voulez et c'est bien que ce soit un médecin. Et et qu'il ait un salaire beaucoup plus important, moi moi je suis pour qu'il y ait davantage de médecins libéraux. Donc j'avais dit ça 5000 euros la coordination dans l'article de mais ça c'est très bien parce que les maisons de santé de toute façon favori cette coordination et il faut aller dans ce sens. je pense aussi que avec les, les CPTS, il faut essayer d'avoir. Ben un accès aux soins. C'est-à-dire. Un accès aux soins non programmés. Et et je pense que c'est possible avec le laisser PTS et je pense que

des gardes à faire et et ça c'est, ça me paraît tout à fait normal. Alors par contre le conventionnement sélectif ce qui était dans l'article cap. Moi je suis aussi favorable. Mais par contre dans l'article 5, je répète que je suis favorable à ce que les médecins qui s'installent en mettent en médecine libérale, hé bien soit favorisé. Je ne suis pas du tout contre les centres de santé. Pas du tout compte, les centres de santé mais je suis favorable à ni contre les médecins salariés mais je suis favorable à ce qu'on favorise les médecins libéraux. Merci. Merci je, mes chers collègues, nous. Monsieur rapporte. Ah oui oui bien sûr.-- Merci madame la présidente. les remarques parce que dans tous les cas on on a lu et on continuera à lire avec intérêt le rapport qui a été réalisé et c'est toujours source d'inspiration pour les débats futurs voilà pour simplement voilà je voulais en tous les cas marqué remercier notre rapporteur tout simplement.-- Bien sûr, ce dernier article 6. J'ai également saisi d'une demande de scrutin public. Allez pour le site, nous le faisons. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Avant, on ne peut pas avoir non plus des crédits de gage qu'on garde pour un autre texte.

La proposition de loi n'est pas adopté et je vais lever la séance et la prochaine séance aura lieu mardi 13 décembre à 9h 30 pour les questions orales. La séance est levée.